La séance est reprise. La parole est à monsieur Henri Cabanel pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci madame la présidente lors du scrutin numéro 155 portant sur la main demain 3937 rectifié mon collègue Bernard filles à l'air souhaitent voter contre. Merci. Merci. Données de votre mise au point et elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. Et maintenant, la parole est à madame la présidente associe pour un rappel au règlement. Merci madame la présidente, mon intervention se fonde sur la le chapitre 14 de notre règlement relatif aux entre autres aux conditions de dépôt des projets de loi. L'article 39 de la Constitution édicte dans son deuxième alinéa ce principe intangible, ce site. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposé sur le bureau de l'une des 2 assemblées. Un avis a donc été rédigé sur ce projet de loi. Le contraire serait a priori anti-constitutionnelle. Vous avez affirmé hier, monsieur le ministre, je vous cite, sur les projets de loi de financement de la Sécurité sociale comme sur les projets de loi de finances. Le Conseil d'État ne rend pas d'avis, il remet au secrétariat général du gouvernement, une note de synthèse. Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer solennellement vos propos d'hier, niant l'existence d'un avis. Ou si s'établit existe. Pouvez-vous concrètement agir pour sa publication rapide afin, cela a été dit à plusieurs reprises par plusieurs collègues afin d'éclairer nos travaux. Quant aux notes que vous évoquez qui selon la presse évoquent l'inconstitutionnalité de votre projet. Je pense. Monsieur le Ministre qu'il serait tout à fait justifiée. Que nous ayons à disposition. C'est notre

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Loi de finances de l'État. Budget, l'État. Loi de financement de la Sécurité sociale. Le Conseil d'État remet au secrétariat général du gouvernement et donc au gouvernement une note sur le projet qui a été soumis. C'est une note avec un certain nombre d'observation. Cette note est à la disposition du. Du secrétariat général du gouvernement. Cette note peut contenir un certain nombre d'appréciation sur les dispositions sur leur recevabilité. Mais ça n'est pas un avis au sens habituel du terme. Je vous confirme un 2ème point madame la présidente. En 2015, le président François Hollande a décidé par une décision orale, cela a été rappelé par je crois. Le président du groupe socialiste hier ou avant-hier que les avis du Conseil d'État et là je parle d'avis accompagnant la publication l'examen en conseil des ministres d'un projet de loi serait rendu public et depuis c'est une doctrine constante que de rende public l'avis du Conseil d'État sur les projets de loi. Il avait été décidé à la même époque par le même président de la République que les notes avec des appréciations des commentaires des évaluations remis par le Conseil d'État gouvernement dans le cadre de son rôle de conseil du gouvernement pour les lois, les lois financières ne serait pas rendu publique je je ne suis pas, vous le savez, président de la République, je n'ai pas autorité pour décider de telles choses. Et donc en l'état, en application de la décision orale prise par le président de la République en exercice en 2015. Les avis du Conseil d'État sur les projets de loi sont rendus publics, les notes rédigées par le Conseil d'État sur les lois financières sont remises. Sans être publié et seul un certain nombre de parlementaires au pied de la fonction de contrôle et de prérogatives particulières peuvent en demander la consultation auprès du secrétariat général du gouvernement. Merci à données de ce rappel au règlement. Alors nous reprenons la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Oui. Madame la présidente au merci à la la présidente mon rappel au règlement, se fonde sur chapitres 14 je ne me. Encore hein. Et je crains que ce ne soit pas forcément le dernier, mes chers collègues. Allez-y même présidente. je ne mettais pas exprimé jusqu'à cet instant sur cette affaire de rapport. Mais l'intérieur l'intervention du ministre que j'ai entendu plusieurs fois. Reconnaissons-lui une certaine constance dans ses réponses me m'amène quand même à réagir, vous dites. Le président Hollande en 2014, a décidé de rendre publics les avis du Conseil d'État sur les projets de loi et les notes du Conseil d'État ne sont pas rendues publiques mais il n'est écrit nulle part que ces notes du Conseil des. As ne peuvent pas être rendu public. Il relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement le vôtre en l'espèce de décider de rendre publique une note qui n'est pas obligatoirement rendue publique. Donc vous jouez sur la nuance entre publicité obligatoire et publicité non obligatoire mais le non-obligatoire n'interdit pas de rendre publique la note. C'est ce que mes collègues vous ont déjà demandé à plusieurs reprises.

Je voudrais comprendre, Monsieur le Ministre, vous vous dites qu'il n'y a pas avis du Conseil d'État. Or dans le dernier Plfss. De 2023. Il y a écrit la Première ministre décrète. Le 1er pour le présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Pour 2023 délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre et donc il s'agit d'un PLFSS avec avis. Mais par ailleurs je vois que notre collègue Savary est présent. Et je me permets de l'interroger puisqu'il est président de la mission de contrôle du PLFSS et je voulais lui demander s'il avait pris connaissance de ce tabou de cette note et s'il serait pas opportun qu'ils nous ont décrive le contenu. Merci. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Je voulais simplement indiquer la madame la présidente Rossignol que. La décision rendue publique, une note du Conseil d'État sur une, sur un texte financier. Par parallélisme des formes, pourraient être pris prise par un président de la République. Ce que je ne suis pas et en en vous disant et en rappelant les règles qui sont fixées depuis la décision orale du président Hollande je dis là ma fidélité à la doctrine qui est la sienne, un peu comme en matière de politique économique. vous plaît. S'il vous plaît. Nous reprenons donc la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Monsieur, monsieur le rapporteur. Vous vouliez. Merci madame la présidente. Effectivement, c'est non pas en tant que rapporteur mais en président en tant que président de l'Amex, soyez assurés que nous avons fait notre travail. J'ai d'ailleurs été étonné que vous ne posez pas la question avant. Mais. Vous vous êtes repris vous être pris, c'est très bien oui. Moi aussi j'ai fait en sorte d'avoir toutes les dispositions. Qui sont. Nécessaires et en tant que président, je peux avoir les mêmes prérogatives. Mais le faire sans forcément de publicité mais de façon et c'est la différence avec l'Assemblée nationale que nous cultivons nous travaillons au fond à l'abri des médias de façon à pouvoir faire en sorte de vous présenter des textes qui ont été travailler différemment, c'est le principe du bicamérisme cette note j'ai pu la consulter, elle, elle contient rien de scandaleux. Elle alerte sur quelques dispositions qui nous avait pas échappé. Quant à leur éventuelle constitutionnalité c'est le travail effectivement on demande à travers ça, donc des dispositions très claires, par exemple par rapport à l'index du senior par rapport à aux cotisations. De. De l'assurance. Agirc-Arrco et transmise le refus en tout cas que le recouvrement des cotisations de l'argile. Se fasse par l'usine safe et et une autre disposition en ce qui concerne la prise en compte des visites médicales qui ne rendent pas directement dans. Effectivement, l'épure d'un PLFSSR. Oui il y a rien d'extraordinaire. Simplement, ce sont des alertes. Tout à fait. Courante et qui ne remettent pas en cause les discussions que nous pouvons avoir au Sénat, merci. Merci madame. Ah pour ce polie pour. Le même article. Rappel au règlement, mais oui oui, je n'avais pas de doutes, Monsieur Savary que vous aviez fait votre travail en tant que président de la messe, mais comment se fait-il que nous ne les ayons pas eu nous, puisque nous sommes à l'Amex. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas remis les notes que vous allez. Que vous êtes allés chercher. Donc pour faire votre travail comment s'est-il que vous nous avez empêché de faire le nôtre puisqu'en tant que membre de l'Amex. Nous n'avons pas eu ces notes. Je ne comprends pas mais je vous rassure Monsieur Savary. Nous allons aller les chercher ses notes puisque vous ne nous les avons pas de vous ne les avait pas remis aux membres de l'Amex. Eh bien nous allons aller les chercher parce que nous sommes aussi vice-, président de la Mecque et que nous pouvons le faire, donc nous irons les chercher. Merci madame de La Gontrie. Merci madame la présidente. C'est sur l'article 19 bis. Ah je crois que ce qui se passe à l'instant est à la fois important et assez grave. Parce que. si l'un de vous est gêné parce que je dis n'est pas obligé de l'écouter. Parce que depuis, nous sommes tous parlementaires ici, donc vous pouvez quand même respecter ceux qui s'expriment.

À plusieurs reprises, a été demandée par plusieurs de nos collègues. Communication de ce qu'a d'abord été présenté comme un avis et qui, aux dires du ministre se. Qualifiait de notes. À plusieurs reprises, nos collègues du groupe écologiste ont réinterroger le gouvernement. Je suis extrêmement frappé et surprise pour ne pas dire choqués. Que le président de l'Amex par ailleurs rapporteur du texte n'ait pas cru devoir préciser. Que justement il était en situation d'avoir eu accès à ce document. Il me semble que le résumé qu'il vient de faire de manière assez désinvolte. Ouais. Et là aussi un problème. Et je demande.

du contenu de la note à laquelle il a eu accès. Étant entendu qu'effectivement les autres membres de cette mission vont sans doute dès demain ou après-demain se procurer cette note puisque vous n'avez pas cru devoir informer les parlementaires de ce travail. Merci Monsieur le Président compta. Oui merci madame la présidente, rappel au règlement sur l'article 19 bis de la même manière, je pense qu'on est quand même face à un problème on peut pas dire monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, qu'on vous a pas demander et redemander depuis l'ouverture. de cette séance et notamment manquait mon collègue Daniel Breuiller de nous transmettre ça cette cette note. Depuis, depuis le début j'entends les explications de de Monsieur le Ministre. Franchement, je veux dire quand on voit ce ce texte qui est demandé par tout le monde qui a priori vous n'avez rien à cacher. C'est ce que vous dites nous avait même dit que on pouvait lire des choses dans les journaux. Et qu'on avait qu'à aller. Lire les journaux pour avoir des informations. Je pense qu'à un moment il faut être sérieux. On est sur un texte sérieux, il me semble que vous pouvez transmettre cette note et puis après. après. Monsieur le. Le rapporteur de la même manière, vous nous avez expliqué vous venez nous expliquer, c'est vrai que ça arrive un peu tard que vous avez eu connaissance de cette note. Moi, je demande la même chose de ce qui a été demandé, c'est qu'est ben une date sur la note peut être hein. En tout cas un une note précise qu'il soit transmis aux membres de la commission et qu'on ait l'ensemble de ses, de ses merci. Madame Lienemann toujours pertinentes. Voilà a posé la question je vous cache pas que j'ai été surpris qu'on ne me la pose pas avant, donc chacun ses prérogatives, chacun ses responsabilités et je pense qu'à travers les dispositions que l'on prend depuis un certain nombre d'années, on monte, bien que nous sommes capables de prendre nos responsabilités.

Alors vous me direz. Qui est la présidente de la commission, le rapport. En général, le président de l'Amex et qui en aucun cas ne doit la rende public. Enfin quand même, c'est comme si vous me porter atteinte. Je ne sais pas moi au secret médical. C'est la même raison et en conséquence je suis tout à fait ouvert d'en parler publiquement, je peux le faire les de façon légale en parler publiquement. Nous pouvons. En discuter si vous le souhaitez, mais en aucun cas cette note ne peut être publié. Telle est la loi. Je respecte la loi et je suis sûr que vous aussi vous êtes dans les mêmes dispositions d'esprit. Merci Monsieur Breuiller. Je pensais qu'il existait dans l'assemblée a une confraternité parlementaire qui aurait permis de renseigner un tout jeune sénateur comme je le suis sur le fait que certains de nos collègues avaient accès à ce sujet mais cet accessoire. Cet accessoire. Ce qui ne l'est pas. Monsieur le rapporteur. Et Monsieur le Ministre, c'est que dans peu de temps, nous allons débattent d'un article de. Dans cette note dit qu'il est probablement inconstitutionnel. Et donc nous allons consacrer du temps sans aucune information des parlementaires ah débattent d'un article qui d'ailleurs a été éliminé par nos collègues de l'Assemblée nationale sans avoir à connaître cet élément, excusez-moi c'est substantiel et c'est un une atteinte à la sincérité de nos débats.

c'était pour continuer la. Solution. Non non non non c'est un rappel au règlement, il faut donner l'article donc chapitres 14. L'article. 9 bis. Voilà. Donc je pense que pardon. que. Que que. Alors, soit monsieur le président de l'Amex. Vous, vous n'avez pas le droit, certes de nous la photocopier, ça nous le savons mais vous pouvez peut être nous la lire. Ça nous évitera un voyage. Parce qu'on va perdre du temps, on a beaucoup de travail ici. Donc. Si vous la lisiez ça serait franchement aussi vite fait. Merci monsieur Chantrel pour un dernier appel. Non, non. Dernière appel qui j'espère aura gain de cause en vertu de 19 bis. Je constate d'ailleurs par rapport à l'appel au règlement de de ma collègue Marie-Pierre de de La Gontrie, vous n'y avait pas répondu à vous a dit justement de pas réponde de manière Cavaliere mais précise sur les éléments qui sont contenues dans ce document pour éclairer les débats. On assiste d'ailleurs depuis le début à une véritable collusion entre le gouvernement et la majorité. Sénatoriale que ça soit sur ces sujets-là comme si il y avait un pacte pour ne pas divulguer des éléments sur sur le projet de réforme pour les parlementaires. Mais qu'est-ce que vous avez à cacher divulguer le nous, on est là pour débattre, on est là pour parler du fond. Donc, parlons du fond et donnez-nous tous les éléments et pas de manière Cavaliere comme vous l'avez fait, mais avec détail et précision pour que le Parlement soit informé comme il se doit, afin de pouvoir justement comme l'a dit très bien dit monsieur brailler. Pour qu'on puisse débattent pleinement de l'article 2 qui viendra après. Monsieur le président Laurent mais c'est le dernier rappel au règlement, merci. Sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, un avis du Conseil d'État. Il y a eu un avis du Conseil d'État. On a le texte. Donc qui le dit. Donc est-ce que sur le PLFSS. Il y a eu celui que nous discutons en ce moment, pourquoi il n'y aurait pas d'avis du Conseil d'État. Et soit disant seulement une note alors qu'il y a habituellement sur chaque PLFSS un avis du Conseil d'État. Vous dites il n'y a pas d'avis sur les sur les PLFSS si il y a un avis sur les PLFSS. Donc il y a quelque chose qui n'est, qui n'est pas très clair et sur lequel nous aimerions la précision. Merci. Merci. Alors nous reprenons la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 dont le Sénat et saisi en application de l'article 47 tirer un alinéa 2 de la Constitution et dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'amendement numéro 3998 rectifié au sein de l'article 1er. L'amendement 3998 a été retiré, passons donc à l'amendement. 4004. Madame ah pour merci madame la présidente. fixant l'obligation obligatoire au régime général c'est un dévoiement même du régime général de la Sécurité sociale. Le qui pourrait désormais intégrer tout travailleur quel que soit leur statut. C'est un pied dans la porte car le gouvernement semble préparer l'opportunité d'élargir à d'autres régimes spéciaux épargnés pour le moment une affiliation au régime général. En tout état de cause rien ne lie empêcherez si ce n'est de revenir devant le Parlement, ce qui ne manquerait pas de faire avec l'assentiment de la droite sénatoriale, cette droite CNS tutorial toujours prompt à donner ses voix à une nouvelle régression sociale si ce n'est pour l'intégration des quelques régimes dits spéciaux qui demeurent à l'issue de cette réforme des retraites peut être le gouvernement envisage-t-il d'intégrer au régime général d'autres risques sociaux toujours couverts par les régimes spéciaux dans une forme de mouvement qui conduirait à se dire en se frottant les mains, les droits à la retraite et après un dernier point suscite notre interrogation mais il n'y a sûrement il y a sûrement une explication, pourquoi ne pas avoir procédé à ce que vous qualifiez comme une précision une précision légistique au moment de l'enterrement du régime spécial. Les nouveaux entrants cheminots. Merci. Alors je vais passer la parole à la commission. Monsieur le rapporteur, madame la rapporteure et avant je signale à l'Assemblée que nous aurons un scrutin public. Merci Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, en fait, en supprimant ces alinéas vous créez un vide juridique pour ces personnels qui sont concernés. Et puis c'est un avis défavorable, parce que c'est contraire à la position de la Commission. Merci. Merci l'avis du gouvernement, même âge, merci. Alors donc j'ai été saisi par donc d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement, l'avis de la commission est défavorable du gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin clos. Résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 339 pour 98 contre 241, le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à 50. 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 4000. 13 ans. Même la présidente Assassi. Même Lienemann. Oui la chers collègues on entre dans le débat sur. Le, le système de retraite des membres du CESE. Alors. D'une manière générale, nous sommes opposés à la remise en cause des régimes spéciaux. Mais dans le cadre du CESE. Je pense qu'il y a une autre préoccupation qui doit être la nôtre.

Nous n'accepterions et la constitution d'ailleurs le prévoit. Pas que ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat voit au système de retraite. Délibérée par une autre instance qu'même en l'occurrence nous pour notre système. Je pense qu'il serait correct. Que le Sénat. Avant toute délibération éventuelle. Pour remettre en cause ce système. Demande au CESE. Quel est son analyse de l'avenir de son système de retraites. Le consulte, c'est pour savoir premièrement si la la même évaluation des risques financiers d'équilibre puisque je rappelle qu'un rapport du du Sénat avait évoqué ce sujet. De s'ils ont des propositions concrètes à faire car comme toutes les assemblées actuelles. Je ne doute pas qu'ils doivent réfléchir à la pertinence de leur système de retraite au regard de ce que nos concitoyens pensent de nous assemblée. Je n'insisterai pas sur notre système à nous nous-mêmes mais en tout cas notre groupe trouve tout à fait inacceptable qu'on n'ait pas eu cette démarche d'avoir d'abord une saisine du CESE sur l'avenir de son système de retraite.

Nous avons eu. Déjà l'occasion de, de l'exprimer. Nous sommes opposés à la fermeture des régimes spéciaux. Ceux-ci correspondent à des conditions de travail particulière et trouvent pleinement leur légitimité aujourd'hui à l'heure où la façon dont on appréhende le travail s'est profondément modifié. Cette volonté de fermer les régimes spéciaux n'obéit à aucune logique ni social ni économique. S'inscrit seulement dans une stratégie de diversion pour tenter de justifier une réforme qui portera préjudice à l'ensemble des salariés en différents de 2 ans l'âge du départ à la retraite c'est pourquoi cet amendement vise à ne pas fermer le régime spécial de retraite du Conseil économique, social et environnemental. Je vous remercie. Merci. Alors. Le 371, madame Ferré. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, cet amendement donc vise à supprimer les alinéas 24 à 27 et 41 de cet article 1er. Qui porte sur le régime spécial du Conseil économique, social et environnemental. Ma collègue leur rappeler. Nous nous opposons à la suppression de ces régimes spéciaux. J'ai envie de vous poser encore et toujours la même question, pourquoi le régime spécial du Conseil économique, social et environnemental. Comment a été opéré le tri entre guillemets entre les régimes spéciaux, je rappelle qu'il y a 42 régimes spéciaux 4 sont donc concernés par cette ce projet de loi. Toutes ces questions restant le suspens depuis que

c'est effectivement la question qui vient tout de suite hein, c'est-à-dire que pourquoi ce régime spécial fait l'objet d'une cible particulière. je ne connais pas le système de régime spécial du CESE. Et je pense que effectivement. Il faut se rallier à la position de Madame Lienemann sur le fait que il faut d'abord consulter l'Assemblée les membres de cette assemblée sur le régime et sur leur leurs critiques sur ce régime là. Et faire en sorte que si on devait y apporter quelques modifications, ce soit à l'Avantage de ses membres. Je vous remercie. Merci. Alors le 509 monsieur Chantrel.

Des alinéas qui vise à fermer le le régime spécial de retraite du du 16. Mais quelque part la la réflexion qu'on pourrait avoir, qui serait peut-être plus large qui est pas liée uniquement à cette à cette réforme des retraites et qui est liée à ces régimes spéciaux. C'est la fameuse question du statut des élus. Je suis sûr que d'ailleurs ça vous intéressera aussi parce que ça nous concerne tous et toutes. Statut des élus bien évidemment aussi pour les élus locaux. Parce qu'on s'aperçoit qu'il a quand même une crise de la vocation importante. Il y a une difficulté à avoir et c'est un fait. Des fois une représentation à l'image de notre pays une mixité justement à l'image de de notre pays. Difficultés, moi je peux en témoigner. Personnellement quand on n'est pas, n'a pas la la protection éventuellement de l'emploi. Qu'on a des carrières hachées. D'ailleurs, qu'on peut aller partout, de pouvoir s'engager s'enfiler après en n'ayant aucune protection éventuelle avec des réinsertion des fois pas évidente. D'ailleurs on a beaucoup d'élus locaux, des fois qu'ont beaucoup de difficultés à se réinsérer. Ça n'est pas forcément valorisé. Je pense qu'on doit vraiment travailler, avoir une réflexion pour faire en sorte, en tout cas de protéger nos élus pour qu'ils puissent s'engager, il faut favoriser l'engagement et c'est pas notre chambre qui va y être opposé, bien au contraire, il faut la favoriser. Il faut travailler le régime des retraites en fait partie. Quand je vous parle de statut de l'élu, c'est parti, c'est lié aussi à pouvoir cotiser pleinement quand on est élu pour pouvoir bénéficier de régimes de retraite. Mais c'est une réflexion, je pense qu'on devrait approfondir pour permettre cette avancée pour la démocratie pour notre pays pour qu'il y ait beaucoup plus de de personnes qui puisse s'engager, d'où qu'elle Vienne. Merci. Alors le 523. Pas défendu. Le 572. Madame de La Gontrie.

Nous arrivons donc au dernier régime que vous avez choisi de sacrifier. Mais nous n'avons toujours pas d'explication quant à vos choix de suppression si ce n'est peut être. De montrer pour l'exemple que vous n'avez pas seulement ciblée les 2 régimes emblématique de la RATP. Il y a des industries électriques et gazières. Qui sont sans doute la vraie cible de votre projet de loi donc pour ce régime du Conseil économique et social environnemental comme pour les précédents, nous souhaitons la suppression des alinéas 27 24 à 27 et 41 qui organise la fermeture de ce régime du CESE. Merci. Alors le 671. Madame Le Houerou. Merci madame la présidente donc par cet amendement. Nous ne demandons le maintien du régime spécial des membres du CESE. Le 16 est composé que d'élus engagés au service de l'intérêt général ils ont des responsabilités dans des syndicats des organisations de jeunesse de coopératives, des organisations représentant les artisans et cetera et ils défendent la protection de la nature et de la biodiversité dans une tribune publiée le 18 janvier, des membres du CESE ont tracé 6 axes de transformation incontournable pour un système de retraite à la hauteur des défis du 21ème siècle, faire contribuer les revenus financiers du capital entré dans une autre relation avec les entreprises pour conforter la cotisation sociale avec par exemple un système de modulation réexaminer tous les dispositifs d'exonération de cotisations sociales patronales qui encouragent souvent les bas salaires et alors quand je lis ces recommandations. Je m'interroge cette réforme inscrite dans un PLFSS rectificatif me semble ne pas y avoir sa place. La réflexion n'est pas abouti et pourquoi ce régime spécial du CESE se retrouve dans une liste de 5 sur 17 de régimes spéciaux, quels sont les critères retenus par le gouvernement pour fermer ces régimes spéciaux en particulier, je n'ai toujours pas compris après de nombreuses heures de discussion. Il n'y a aucune urgence à inscrire cet article qui mériterait. Que nous consultions le CESE sur ce sujet comme sur les autres éléments de d'une réforme de de retraite abouti. Merci. Alors le 700. Madame la truc ce compta. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à ne pas supprimer le régime spécial du CESE. Dans d'autres ici dans l'histoire de notre République, le Conseil économique et social occupe une place particulière, il y a une forme de provocation politique grave en touchant en touchant au régime spécial de ses salariés sans qu'il soit consulté, qu'il délibère le Conseil économique et social est né de la résistance du travail de conviction des syndicalistes résistance et sur son modèle qu'en 1957 les pères fondateurs de l'Europe ont créé via le traité de Rome, un conseil économique et social européen. Elle les travaux du CESE contribue à éclairer les citoyens les législateurs que nous sommes sur tous les grands sujets sociaux, environnementaux. L'actuel président de la République n'aime pas le 16. De manière générale, il n'apprécie guère l'indépendance des organisations syndicales, des associations et toutes les autres libre expression de la société civile aussi dès 2017 le bruit avait couru de sa suppression pure et simple. Et de la dispersion de ses agents finalement pour tenter de le marginaliser, il a été beaucoup transformée réduit dans le nombre de ses membres et donc s'opposer à la suppression du régime spécial du Conseil économique, social et environnemental, c'est aussi s'opposer à son affaiblissement. Ne touchons pas à cette assemblée délibérative essentiel à notre République et à notre démocratie. Merci. Alors le 731 le 813 le 826 et le 866 ne sont pas défendus le 901 Monsieur Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, chers collègues. Je me rallie à ce qu'a.

Nono. Nono, madame, ce n'est pas un rappel au règlement. Je vous dis que on demande. La suppression de ces alinéas. Ne pas remettre en cause le régime de retraite de ces parce que je pense qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité. C'est pas un appel au règlement de dire que premièrement il faut une consultation. Deuxièmement, l'article 70 de la 71 dit la composition du conseil et ses règles de fonctionnement relève d'une loi organique. Parce que je suis clair. J'estime moi que le régime de retraite, c'est le mode de fonctionnement du CESE et là on le modifie, par une loi de financement, voilà c'est pourquoi je demande à soutenir l'amendement de suppression de.

Je crois qu'il est assez bien défendu par les interventions précédentes. En toute hypothèse, en ce qui me concerne, bien sûr je. Soutiendrai les. Amendements. Qui permettent de maintenir ce dispositif dans le même esprit que nous l'avons fait depuis le début de l'examen de cet article. Nous considérons que les régimes spéciaux ne sont pas le signe de privilèges mais tout simplement une adaptation de notre réglementation et de notre législation a des particularités de certains métiers et de certains statuts qu'il s'agisse. Du fonctionnement institutionnel des organismes dans lesquels. Les. Salariés. S'inscrivent qu'il s'agisse de particularités liées aux conditions de travail propres à certains métiers, dans tous les cas il n'y a pas de motif à uniformiser de façon. Aveugle et systématique. L'ensemble des dispositifs relatifs à la retraite parce qu'il y a plein de façons d'exercer sa responsabilité professionnelle et donc nous proposons le maintien de ce régime particulier. Merci. Alors le 1155. Mesdames Lubin. Le 16 est composé d'élus qui sont engagées en règle générale, dans un certain nombre. D'associations ou de structures qui sont dévolus à l'intérêt général. Ils ont des responsabilités dans des syndicats des organisations de jeunesse, des coopératives et ils défendent. Un grand nombre de nobles causes, bref ce sont des gens engagés un petit peu comme les élus dont j'ai entendu parler tout à l'heure.

Concernent finalement peu de gens et nous nous demandons bien pourquoi on va les chercher sur ce projet de loi. Une fois de plus, nous avons l'impression que. Deux ou trois régimes un petit peu particulier ont été mis dans le lot pour pouvoir jouer, on va dire. Groupés avec des régimes comme ceux des gaziers ou de la RATP. Que vous avez envie de faire sauter si je puis m'exprimer ainsi, depuis un moment. Donc bon nous demandons effectivement la suppression de ces alinéas nous ne nous considérons que ce projet de loi de finances qui est fait uniquement pour reporter l'âge de la retraite de 2 ans et clairement, pour faire économiser de l'argent aux finances de l'État ne devrait pas contrevenir à l'avenir d'un certain nombre de salariés de ce pays qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas de privilège particulier et dont les systèmes de retraite ne nécessitent pas. Comment dire que l'on, que l'on aille, ah d'abord qui n'aggravent pas la situation des régimes de retraite, en règle générale, il ne nécessite pas. Qu'on aille leur empoisonner la vie. dit ce n'est pas soutenu le 1249 madame Jasmin. Merci madame la présidente. Je suis pour le maintien du régime spécial des retraites du CESE. On ne peut pas s'attaquer aux régimes des retraites du 16h dans un PLFSS rectificatif ça déjà été dit. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait le choix de perturber un système démocratique, pour le rendre, je ne sais même pas comment le qualifier, parce que dans une vraie démocratie, hé bien on ne s'attaque pas à ce qui fonctionne, on crée des dysfonctionnements. Et je crois que ce que vous proposez aujourd'hui monsieur le ministre a et c'est que l'ensemble du gouvernement en 2017. Hé bien, rappelez-vous. Vous avez voulu. Également éliminé le Sénat et peut être l'ensemble des personnes qui travaillent ici au Sénat, et comme vous avez bien compris que ce ne serait pas possible parce que nous défendions la démocratie vous vous attaquez. Au 16h. Et vous voulez faire disparaître cette instance qui joue un rôle très important. Pour les Français. Pour la société et pour la démocratie. Merci madame la présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre. Toujours dans votre logique qui confine à l'obsession de destruction des statuts ou des dispositifs tant soit peu protecteur. Vous voulez être mettre maintenant enfin au régime spécial du CESE. Rien ne justifie cette suppression. Son existence participent de l'attractivité des métiers de cette institution de la République qu'est le 16 et je rappelle ici les contributions importantes. De cette. Chambre à la démocratie sociale et participative. Dans notre pays a besoin pour évoluer dans tous les domaines de la vie de la nation, la qualité de travail des fois actionnaire du CESE est à cet égard remarquables, il faut la préserver. L'article 1er la sacrifie. Cette suppression est aussi le nouvelle démonstration du peu de considération que vous portez avec le président de la République au corps intermédiaires. Nous pensons le contraire hein à l'égard du CESE et des fonctionnaires concernés et nous opposerons et nous nous opposerons à la suppression de ce régime de retraite des fonctionnaires du CESE en rejetant l'article 1er. Merci le 1319 madame Préville. et à cette heures toujours une stigmatisation d'un régime spécial qui est injustifiée. Le nivellement par le bas n'est pas une réforme, c'est une régression. À cela s'ajoute la question très épineuse s'agissant d'une assemblée délibérante comme l'a rappelé notre collègue Marie-Noëlle Lienemann cela paraît pour le moins singulier de statuer sur ce sur ce régime. Car la question reste toujours entières à ce, à cette heure-ci. Pourquoi ce choix. L'engagement des membres du Conseil économique, social et environnemental est-il à questionner. Leurs recommandations, leurs travaux, leurs préconisations pose-t-elle problème par contre on ne peut nier le travail de fond qui est menée. Si cher collègue. Le 1343 n'ait pas défendu le 1376 Monsieur Bourgi. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À l'instar de mes collègues sont intervenus. Juste avant, moi je voudrais insister sur l'importance de garder le régime spécial du CESE. Monsieur le Ministre, je m'adresse à vous, il y a plusieurs dizaines de régimes spéciaux en France. Pour quelle raison vous en avez choisi quelques-uns parmi tant d'autres. Quelles sont les motivations budgétaire et financière. Quelles sont les motivations idéologiques, politiques, quelles sont les motivations juridiques. Nous avons besoin d'être éclairé. Je ne voudrais pas que derrière le choix de ces régimes spéciaux, il puisse y avoir une suspicion d'un délit de sale gueule. Je ne voudrais pas que derrière le choix de ces régimes spéciaux. Un acte de défiance politique qui a été posée par votre gouvernement. Deuxième observation qui s'adresse cette fois-ci à vous mais aussi à nos collègues de la majorité sénatoriale. Le CESE. Ce n'est pas n'importe quel organisme le 16. Est une instance est une chambre importante pour la démocratie nationale. À l'instar de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pourquoi cautionner nous ici la remise en cause du régime spécial du CESE. Pourquoi ce qui concerne le 16 ne s'appliquerait qu'ils pas demain à l'Assemblée ou au Sénat, vous l'avez compris, mes chers collègues. Il y a ici un acte politique. Je vous invite tous et toutes au sursaut parce que le sale coup que le gouvernement porte contre le 16 aujourd'hui. Il pourrait le porter demain contre l'Assemblée au contre le Sénat concernant les régimes autonomes mais aussi sur d'autres sujets il me semble qu'il nous appartient de faire preuve de solidarité avec les autres chambres qui sont saisis qui sont consultés comme le gouvernement et le président de la République vient de le faire sur la fin de vie par exemple, on ne peut pas louer en permanence la qualité scientifique, l'expertise des travaux du CESE et venir réserver un sale coup à cette chambre. Si alors le 1409 1439 1507 ne sont pas défendus 1546 Madame Monnier. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Donc cet amendement vise le maintien du régime spécial de retraite du Conseil économique, social et environnemental. La méthode interroge pourquoi procéder de cette manière à la suppression de ce régime propre à notre 3ème assemblée. Je rejoins mes collègues sur le fait que c'était certainement parmi tous les régimes spéciaux qui existe de pouvoir enrobé la suppression du régime spécial de la RATP. a des l'industrie électrique et gazéifié. Si on regarde depuis 2017 à plusieurs reprises, le président a fait aussi part de son manque de considération du CESE. On peut considérer que le grand débat la Convention citoyenne pour le climat. Plus récemment le lancement du conseil de la refondation sont ainsi autant d'exemples où le gouvernement a voulu passer outre cette instance pourtant elle est représentative de forces vives économiques, associatives et syndicales du pays 175 élus engagés au service de l'intérêt général. c'est sûr que la suppression par ce véhicule législatif du régime de retraite propre au CESE constitue une autre preuve du manque de considération du gouvernement à son égard et je reprends aussi les propos de mon collègue qui s'exprimer jusqu'à 20 mois à savoir pourquoi est-ce qu'on devrait faire une exception de ce qui se passe au Sénat et pourquoi on ne devrait pas s'interroger sur le fonctionnement de notre propre caisse de retraite. Alors le 1595 n'est pas soutenu 1625 madame Pumerole. Oui merci madame la présidente. Une nouvelle fois le gouvernement semble assimiler les régimes spéciaux à des privilèges et souhaite ainsi les supprimer pour motif de soi-disant équité. Comme mes collègues, je me pose la question. Pourquoi cette mesure qui et comment la décider comment a été fait, le choix entre les. Régimes spéciaux supprimés et ceux qui seront conservés puisque seuls 5 régimes spéciaux représentant quelque 350.000 travailleurs au total sont concernés par la réforme. Il semble bien quand même que dans le cas du CESE ce soir pour masquer la disparition. Souhaiter que vous souhaitez du régime de la RATP et des IEG. Vous nous avez parlé d'équité, là on a du mal quand même à y voir clair. Quelle est votre logique. Où est la cohérence. En réalité, cette suppression à la carte né qu'injustice et elle traduit votre volonté de détruire les systèmes sociaux protecteurs. Je vous propose donc par cet amendement de ne pas fermer le régime spécial des retraites du CESE. Merci. Alors le 1655 n'ait pas défendu 1696 Monsieur le comte. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues oui cette disposition dans le projet de loi est assez étonnante. Assez étonnant parce qu'il s'agit de la 3ème assemblée constitutionnelle de la République assez étonnant aussi puisque, à l'été 2020, nous avons voté une réforme du Conseil économique, social et environnemental devant faire de ce conseil revue. Le Carrefour des consultations citoyennes. Et puis. Emmanuel Macron a été réélu et finalement il a décidé que c'était probablement plus important que cette réforme faite en 2020 n'avait aucun sens et il a lancé le Conseil national de la refondation finalement en prétendant faire de cette manière d'autres consultations citoyennes en passant au-delà et par dessus les représentants de la société civile qui était. Au Conseil économique, social et environnemental. Alors c'est vrai que on s'est demandé on se demande pourquoi cette réforme a été faite en en août 2020. Si 2 années après finalement le président de la République et le gouvernement ont décidé de faire ailleurs les consultations citoyennes sans s'occuper des corps intermédiaires. Mais au-delà de cela, il est effectivement comme Marie-Noëlle Lienemann le rappeler étonnant que pour le régime de retraite d'une assemblée constitutionnelle. Cette assemblée ne soient pas consultés. Et. La réforme de 2020, elle a été portée par une loi organique et je m'interroge sur une question comme l'a interrogé comme nous a interrogé Monsieur. Notre collègue Victorin Lurel et et c'est une question que je pose à nos rapporteurs que je pose à Monsieur le Ministre, je serais assez étonné. Que le régime de retraite d'une assemblée de la République qui se réforme par loi organique puisse passer par un PLFSS et pas par une loi organique, comme la réforme de la retraite des magistrats de l'ordre judiciaire par exemple ça me semblerait logique et je vous interroge sur la dit la capacité de mettre cette disposition dans le PLFSS sans risque. Merci. Alors 1752 1794 1822 1849 ne sont pas soutenues. Passons. 1995. Même la présidente Rossignol. Merci madame la présidente. Je pense que il faut qu'on aborde cette affaire avec sérieux et attention. Pas tant. Sur la question en tant que telle, du régime spécial du CESE. Mais de ce que signifie le fait que, à cet instant. À la demande du gouvernement nous puissions mettre fin à un régime de retraite d'une des trois assemblées constitutionnelles de ce pays, c'est ça le sujet. Et que nous le fassions sans eux. En fait il y aurait des assemblées. Nous sommes 3 hein, assemblée nationale, Sénat. 16. Il y aurait des assemblées qui serait. Capable et qui revendiquerait la possibilité de faire évoluer elles-mêmes leur régime de retraite. Et d'autres qui seraient soumises à un PLFSS dans lequel au milieu de dans dans un, dans, dans l'enthousiasme du gouvernement, de sa suppression des régimes spéciaux, on passerait celui d'une absence d'une assemblée constitutionnelle. C'est pas une mince affaire. Mes chers collègues, d'autant que par le passé, le CESE a déjà procédé à un certain nombre de réformes de ses prestations en 2013 parce que nous savons tous qu'il y a un problème de financement de ce régime. Tout le monde a dû dire le rapport de la. Cour des comptes dans le gouvernement a du goût ça inspirer avec gourmandise j'imagine d'ailleurs hein mais en 2013, ils ont déjà diminué par 2. Niveau des pensions. Augmenter les cotisations pris toute une série de mesures pour assainir le régime. Ils l'ont fait eux-mêmes ça veut dire qu'en 2013 il était capable de prendre des mesures pour assainir les et l'équilibre de leur régime mais qu'en 2023 il y aurait besoin d'une intervention du gouvernement de l'exécutif pour assainir et mettre fin à un régime qui le régime d'une assemblée parlementaire. Chers collègues, réfléchissez bien ce que vous êtes en train de faire. Merci. Le 2074 n'est pas soutenu le 2262 Madame Espagnac.

Madame Cohen. Je crois que c'est Madame Cohen. Merci madame la présidente, les régimes spéciaux, donc qui sont t'attaquer à travers cet article 1er ont ont été largement réformé dans une logique de nivellement par le bas. Nous l'avons dit à plusieurs reprises et cette à cette logique que nous nous opposons, vous l'aurez compris, vous nous dites que les régimes spéciaux sont vécus comme une injustice profonde que la réforme sur un instrument d'égalité qui mettrait fin des privilèges insupportable. De quelques profiteurs évidemment nous vous avons répondu depuis le départ de notre discussion que, pour nous, c'est une autre conception, ce sont. Des régimes, au contraire pionnier qui devrait tirer l'ensemble de notre système de retraite vers le haut et non pas donc être supprimés. Le président de la République en appelle au bon sens des travailleurs et des travailleuses pour donc en fait travailler toujours plus et plus longtemps mais où est le bon sens. Mes chers collègues. Lorsque l'on sait que les ouvriers ont une espérance de vie qui est de 6. IV inférieure à celle des cadres. Ou est le bon sens lorsque l'on sait que 25% des hommes et 13% des femmes faisant partie des 5% des plus pauvres meurent avant 62 ans. Où est le bon sens pour quand tu pour beaucoup les dernières années de travail avant la retraite sont souvent rythmé par des difficultés de santé. Je vous rappelle que 14% des ouvriers ont un fort niveau d'incapacité physique dès leurs premières années de retraite où elle bon sens lorsque vous condamnez les travailleurs les plus âgés en fait à beaucoup de précarité et une difficulté à joindre les 2 bouts si je puis m'exprimer ainsi. Car ne nous y trompons pas, les travaux économiques menées sur le passage de la retraite de 60 à 62 ans ont montré qu'il n'y a aucun effet vertueux favorisant l'emploi des seniors en 2019 à 61 ans, un quart des employées et un tiers des ouvriers n'étaient ainsi ni en emploi, ni en retraite votre réforme aura pour principal effet d'allonger encore les périodes de non-emploi avant la retraite pour les personnes concernées. C'est donc le sens de notre amendement. Merci. Il est défendu madame la présidente. Merci le 4025. Il est défendu. Merci.

Oui madame la présidente, notre amendement vise à remettre en cause le détricotage. De notre système de retraite. Mais vous vous en doutiez sans doute la alinéa 35 de l'article 1er amène des modifications conséquentes, notamment pour les professeurs des écoles et documentalistes des études des établissements excusez-moi privé alors évidemment lorsqu'il s'agit de vous attaquer au travail aux travailleurs des établissements. Vous êtes tous rendez-. Vous, vous le savez, nous aimerions que l'école publique et les enseignants qui ont la mission soit suffisamment doté et même aussi bien doté que les établissements privés les établissements publics devrait même selon nous pouvoir bénéficier de dotations supplémentaires au regard des élèves qui en bénéficient et dans un souci d'attractivité pour garantir une mixité que vous contrecarrer cette attractivité ne peut toutefois passer par une atteinte au régime de retraite des enseignants qui ne servirait ni l'enseignement privé, ni l'enseignement public et qui au fond contribuera à dégrader encore un peu plus l'ensemble de l'éducation nationale. C'est pourtant un sujet l'éducation nationale qui est régulièrement brandie comme une priorité par le gouvernement, c'est d'ailleurs ce qui devient inquiétant dans la bouche du gouvernement une priorité est en fait une cible pour ne pas dire une proie. Alors ne faites pas des retraites votre priorité ni la retraite des enseignants ni la retraite de qui que ce soit ne touchez à rien comme vous savez le faire pour les profits qui s'envole. Merci alors de 2746 même Lubin. Et le 2749. Défendu aussi. Je vais donc demander à la vie de Madame la rapporteure. Oui merci madame la présidente. À l'heure sur l'ensemble des amendements qui concerne le le Conseil économique, social et environnemental. Tout d'abord quelques précisions. Les membres du CESE ne sont pas des élus. Ce sont des membres désigner des représentants sociaux du patronat, des syndicats et. Du monde associatif. Donc ça c'est très important déjà de le savoir et ce n'est pas un service public il y a pas séparation des pouvoirs, tels que l'on, on la rentre. Comment ici au Sénat, donc c'est bien une différenciation qu'il faut faire ensuite pourquoi. On on s'est aussi penché sur ce régime spécial, d'une part parce que les cotisations salariales, c'est à peu près un million neuf des cotisations patronales, c'est 2 millions, 9 environ le double et par contre la contribution d'équilibre de l'État, c'est 5,4 millions, donc on voit bien qu'il y a. Une vraie dichotomie entre 175 membres et puis les 800 pensionnés. Et donc c'est pour cette raison que nous avons choisi. De de mettre fin à ce régime. De de de retraite pour le 16 et puis il y a les autres amendements qui ont été proposés. C'est un avis défavorable pour l'ensemble de ces amendements. ensuite il y a les amendements de 4019 à 4106. C'est un avis défavorable. Et puis sur le 2746 est aussi un avis défavorable, parce que c'est la même. Réponse que tout à l'heure en fait ça crée un vide juridique pour le personnel concerné. Et puis. Pour le dernier le 2749 c'est un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. C'est vrai que les les amendements que nous. Examinerons la sont de nature différente puisque les tous premiers concernés l'affiliation au régime général de l'assurance vieillesse des salariés actuellement. Qui aurait dû être actuellement rattaché à un régime spécial. Madame la rapporteure là dit et l'adoption de ces amendements et la suppression des alinéas concernés crée un vide juridique est préjudiciable pour les salariés en question qui ne serait plus affiliés au régime général au régime spécial pardon après le 1er septembre mais qui ne pourrait, du fait de la suppression de l'alinéa être affiliés au régime général pour en venir au régime spécial du, du Conseil économique, social et environnemental et et répondre à quelques-unes des interventions des interrogations qui ont été qui ont été soumis. Est-ce que le Parlement est fondé à réviser et réformer le régime spécial des membres du CESE. La réponse est oui, oui parce que le régime de retraite des membres du CESE est un gym qui est défini par une loi ordinaire du 10 juillet 1957 et cette loi ordinaire du 18.957 a donné lieu à un décret d'application en 1959, décret qui a été modifié par un autre décret de 2017. Et lorsque le Parlement a été saisi il y a maintenant 4 ans, du projet de loi visant à créer un système universel de retraite. Ce projet de loi était accompagné Nasreen Davy qui précisé que le Parlement était fondé dans le cas d'une loi ordinaire, que ce soit une loi ordinaire ou une loi de finances, nous sommes sur le même véhicule juridique à réformer le véhicule le le régime de de retraite des membres du CESE et il précisait même que la comparaison avec le régime de retraite des membres du Sénat ou des membres de l'Assemblée nationale ne tenait pas du fait des caractéristiques de rémunération et de désignation des des membres du CESE. La 2ème, chose que je voulais souligner parce que un certain nombre des sénateurs qui ont défendu ces amendements ont. Évoqué la situation des salariés du CESE. Les salariés du CESE ne sont absolument pas concernés par les alinéas les Alina que vous voulez supprimer les seuls qui sont concernés sont les membres, les conseillers du CESE. Les les salariés du CESE, pour la plupart d'entre eux. Sont des fonctionnaires en détachement ou mise à disposition par leur administration d'origine et donc affiliés au régime de. D'assurance-retraite de leur administration d'origine, il y a un certain nombre de contractuels, mais dans ce cas-là c'est contractuels sont rattachés à la Cnracl ou à l'Ircantec et Ircantec pardon et donc il n'y a pas de difficulté particulière, mais je le répète ces Alina ne concerne que les conseillers du CESE et ça me donne l'occasion de dire que après. L'adoption de cette réforme si le Parlement en décide ainsi. Le nouveau régime d'assurance vieillesse des conseillers du CESE relèvera d'ailleurs de l'Ircantec. Ce qui souligne le lien avec la mission d'intérêt public qui est, qui est la leur. Voilà ce que je voulais dire madame la présidente madame la rapporteure générale a évoqué le, le déséquilibre, même si les sommes sont moins importantes que pour d'autres régimes que nous avons évoqué mais il y a un déséquilibre avec. 175 cotisants pour environ 800 pensionnés aujourd'hui et la nécessité d'une subvention d'équilibre à hauteur de 5 millions quatre par. Merci. Alors sur l'amendement 4013 je suis saisi d'un scrutin public. Donc. Je me demande, il y a des explications sur cet amendement parce que j'ai, j'avais compris que vous étiez plutôt inscrit sur la liste des amendements suivants.

Oui sur cet. Amendement je souhaite faire une explication de vote. Je considère que la l'explication que vient de nous donner Monsieur le Ministre ne retire en rien la. Revendication d'une consultation du du Conseil économique et social en tant que telle, qu'il s'agisse de ses salariés ou qu'il s'agisse de ses membres dans tous les cas et singulièrement s'il s'agit de ses membres, peut-être plus encore que si il s'agissait d'agents salariés ça justifie parfaitement que nous interrogions cet organisme sur le point de savoir quel est son avis concernant la réforme du dispositif de retraite. Merci. Comme l'a dit Monsieur le Ministre, je veux bien le croire sur le fait que le Parlement puisse délibérer sur le système de retraite du CESE. Mais il y a entre l'obligation légale la possibilité légale et la manière de créer des Liens entre des assemblées qui par ailleurs existe dans la constitution. Il y a quand même une question de forme. Qu'au bout du dispositif. On puisse juger après avoir entendu le CESE. Après lui avoir demandé comment il comptait faire face au déséquilibre entre le nombre de cotisants. Et le nombre de bénéficiaires. On soit amené à délibérer. Ne meurt, t'aurais pas forcément. Ce que je trouve tout à fait inacceptable. Et pour le moins cavalier. C'est que le Sénat n'ait pas pris soin. De demander son avis à l'assemblée. Du CESE. Une assemblée où il y a essentiellement les partenaires sociaux. Grandes associations les forces vives de la nation. Alors je sais qu'il est de bon ton chez certains. De mépriser ces corps intermédiaires. Je crois que ça procède d'ailleurs d'une des fragilités actuelles de notre démocratie. Et du rapport que les Français ont à la vie politique et sociale. Je considère donc au-delà de l'obligation légale ou la possibilité légale. L'acte politique du Sénat n'est pas responsable car vous savez, chers collègues. En d'autres temps notre ses nappes de mis en cause. Et le populisme ambiant. Peut trouver des échos. Soyons nous très respectueux de toutes les institutions, notamment quand elle représente les forces vives de la nation.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Le ministre vient de nous déclarer. Que le Parlement peut légiférer, bien sûr, mais qu'il y avait une loi ordinaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal, enfin j'ai entendu une loi de 57 et les décrets d'application. 2017. Bon une loi ordinaire. Moi je persiste et je signe, cette loi n'a pas fait l'objet d'une QPC. Que je dis c'est par loi organique, il faut le faire. Article 71 de la Constitution la présidente à penser que parce que j'avais le règlement mais que c'était un arrêt rappel au règlement non le fondement même Marine Lionel. Parole de forme, il faut consulter ouvrir bien sûr c'est important la forme en démocratie mais là c'est un problème de fond. Je dis qu'il y a un problème d'inconstitutionnalité que le texte qui a été pris et inconstitutionnelle et qui fait l'objet d'un recours d'une question prioritaire de constitutionnalité, on aura un pour la 2ème point où il faut de cette fois-ci de manière idéologique et philosophique voter contre ça. Le président de la République a voulu affaiblir le 16, il a voulu affaiblir pour les corps intermédiaires, il s'était institué en. Conducator hier le leader Maximo. Il ne faut pas qu'il y ait de corps intermédiaires et le sommet des corps intermédiaires, c'est bien le 16 l'affaiblir le diminuer au lieu de l'augmenter est une atteinte à la démocratie à la Constitution. Mais si. Alors donc nous allons faire le scrutin public. Il a été demandé par le groupe CRCE. Sur l'amendement donc numéro 4013 hein. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement aussi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Un résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 339 pour 98 contre 241. Le Sénat. Pas adopté.

Merci madame la présidente, monsieur Ministre, mes chers collègues d'abord. Je vous remercie Monsieur le Ministre des éléments qu'il a pu nous donner Ne sont en rien une certitude mais qui je peux comprendre que sur le faisceau d'informations qui nous donne. Il. Peut raisonnablement penser que c'est jouable de cette manière. Mais c'est vrai que reste l'article 71 de la Constitution. Qui. Interroge et qui laisse finalement compte tenu des dates qui nous ont été donnés. Par Monsieur le Ministre, laisse quand même une incertitude juridique assez forte sur le sujet qui qui méritera finalement d'être pris en pris en compte dans les recours qui pourraient être. Déposées mais à la limite, peu importe. À ce stade. Ce. Cette cette interrogation qui sera tranché le moment venu. Lors de l'examen des recours qui pourraient être déposées. La question les politique. La question est de savoir si. Une assemblée en l'occurrence le Sénat peut décider. Pour. L'assemblée une Assemblée constitutionnelle autre sans avoir même recueilli son avis. Et nous ne considérons pas dans cette partie de l'hémicycle, que compte tenu de l'importance du CESE il soit opportun de décider sur ce type de décision de sur ce type de choses sans avoir l'avis du Conseil économique, social et en du Rwanda. Nous considérons qu'il n'est pas raisonnable de le faire

Oui je voulais expliquer un vote favorable pour l'amendement 2746. Rectifié qui vise à ne pas affiliés des populations très éloignées du salariat. Les loueurs de meublés vendeur de bien sur des plateformes au régime complémentaire complémentaire cet article 1er du projet de loi modifie l'article L. 921 tirer 1 du code de la Sécurité sociale relatif au Champ d'application des institutions de retraite complémentaire pour tenir compte de la filiation des salariés de régimes spéciaux au régime général et complémentaire donc à compter du 1er septembre 2023, la rédaction proposée par le projet de loi aboutit à affiliés à ces institutions, toutes les personnes relevant de l'article L 311 de du code de la sécurité sociale et notamment par toutes les populations visées L 311 tirer 3 du même code. Or, certaines de ces populations étant très éloigné du salariat. Les loueurs de meublés, les vendeurs de biens sur des plateformes type Le Bon Coin ne relèvent pas du régime Agirc Arrco sur décision des partis partenaires sociaux gestionnaires de ce régime. La rédaction du projet de loi aboutirait à faire adhérer obligatoirement ces populations aux régimes Agirc-Arrco. Je soutiens donc cet amendement qui propose de ne pas modifier l'article en question sa rédaction a tenu. Permettant de viser tous les salariés, y compris ceux relevant aujourd'hui des régimes spéciaux et c'est un, un, un amendement qui a été travaillé avec l'Agirc Arrco. Merci madame la présidente, moi je crois vraiment, j'ai le Roddick. Là on a un paquet cadeau et on a des régimes qui n'ont rien à voir d'un côté, la RATP et Liegey ou c'est vraiment une. C'est une pression sur. Le partage des richesses là qui est en jeu, c'est une dérégulation du travail, une une pression sur le salaire socialisé donc sur le partage des richesses et toute la loi d'ailleurs

Les cinq sur les 17 je ne sais pas si on fait partie des 17 là on se demande pour. Quoi et ça a été long longuement dit. Il est évident quand même que s'agissant de la 3ème. Chambre de la République il convient quand même ils ont changé leur régime en 2013 ou 2015, les dates sont un peu imprécise. Toujours est-il qu'à l'évaluation de ce changement. Pourquoi à l'époque c'est eux qui l'ont fait et pourquoi maintenant on. veut prendre la main et effectivement là il y a peut-être. Une conception des des corps intermédiaires et une prise de pouvoir un petit peu sur cette chambre donc. Nous, nous voterons. Pour cette suppression, ne faisons pas l'amalgame, quand même, entre ce qu'il a dans votre paquet cadeau hein et qui n'a qui a des objectifs et des motivations je pense très différentes. Merci madame briqué. Merci madame la présidente. Mes chers collègues. Lors de nos débats, beaucoup de propos. Souhaiter revaloriser les pensions des femmes et où. Et ou réduire l'écart entre celle-ci et et celle des hommes à ce titre-, les régimes spéciaux spéciaux marque une une réelle différence. Les écarts de pensions entre les hommes et les femmes sont relativement réduits dans la fonction publique et dans les, dans les régimes spéciaux, alors qu'ils sont plus importants dans le secteur privé notamment parmi les non salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes sur le Champ des monopoles nationaux à carrière complète est en 2020 de 87% pour les fonctionnaires civils d'État et pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et de 82% pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 71% pour les salariés relevant du régime général et 63% pour les non-salariés plutôt que de hein de fermer hein c'est un c'est régimes il vaudrait mieux les conforter, car il marque une réelle avancée au CESE, comme pour les autres régimes spéciaux. Je vous remercie,

De supprimer le régime spécial des membres du Conseil économique, social et environnemental, comme il le propose soit sur. Pour le régime spécial des des agents des industries. Électriques et gazières que nous avons examiné précédemment. Dans les 2 cas il s'agit d'actes politiques qui remettent en cause à la fois les fondements de notre souveraineté et de notre démocratie. La suppression du régime spécial des industries du gaz et d'électricité s'inspire d'une philosophie libérale qui porte une logique de privatisation et de dérégulation, d'un secteur pourtant essentiels à la souveraineté de notre pays. Parallèlement, donc le gouvernement en proposant de supprimer le régime spécial du Conseil économique, social et environnemental, il s'attaque à ce qui représente un corps intermédiaires. Dont le président n'a pas encore réussi à comprendre, à la fois l'importance et la manière de travailler avec cette institution et comme les autres corps intermédiaires. Et apparaît donc essentiel de s'opposer à cette surpression d'autant que la procédure suivie. Si elle a éventuellement légal voire constitutionnel en tout cas pose le problème de la légitimité à agir de cette manière sans consultation dès lors je soutiendrai les amendements qui concerne la suppression de cette suppression. Alors. Bien évidemment. Je défends ces amendements. Mais Monsieur le Ministre, je viens de lire une à une interview à paraître dans Le Parisien de demain. Ou vous dites. La réforme des retraites ne fera pas de perdants. Liste ici non exhaustive des situations dans lesquelles les personnes seront objectivement perdante à la réforme. Si comme vous on ne considère comme perdante que les personnes de la pension baisse il y aura bien des. Perdantes et des perdants. Les personnes qui, sans réforme aurait bénéficié d'une surcote parce qu'elles ont choisi de travailler au-delà de l'âge du taux plein. Venez leur surcote. Annuler ou diminuer jusqu'à 10 points de pourcentage du fait de la réforme. Avec le passage accéléré à 43 annuités. Je vous donne un autre exemple, les personnes nées avant 1974 pourraient voir leur pension baisser. Notamment si elle ne décale pas leur départ. Mais au-delà du seul montant de pension c'est principalement par le décalage de l'art de de l'âge de départ que la réforme fait des perdants et surtout majoritairement des perdantes. Exemple, une personne fonctionnaire né en 1963 qui devait partir dans 2 ans à taux plein à 62 ans, devra partir dans 2 ans et demi pour la même pension. Et des cas comme ça, j'en ai d'État malheureusement mon temps de parole ne me permet pas de tous les exposés mais un autre exemple, début de carrière à 18 ans sans interruption de départ avant réforme. 62 ans après réforme, 63 ans, des cas comme ça on en a à la pelle. Donc arrêtez les mensonges et retirer cette réforme injuste qui ne fait que des perdants. Merci monsieur Chantrel, je voulais juste vous souligner que là nous étions sur les. L'amendement 240 346 à 2262 et donc là nous étions dans des explications de vote, je vous remercie. Donc je mets aux voix donc ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour.

C'est un rappel au règlement. Au titre de l'article 19 bis B. Depuis hier, j'ai à sept ou huit reprises. Voire plus demander la publication de l'avis du Conseil d'État. Chers collègues. Chers collègues, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est important, je vous demande. s'il vous plaît. C'est monsieur Breuiller qui a la parole. Merci. Donc j'ai demandé à 7 ou 8 reprises la transmission de cet avis. Mes collègues sur tous les bancs de la gauche, l'ont demandé. Marie-. Pierre de La Gontrie. Le président Laurent on re-insister sur ce sujet. On m'a répondu avec un peu de condescendance, que je n'ai pas osé prendre pour du mépris qu'il n'y avait pas d'avis du Conseil d'État. Alors je m'interroge, je l'avais dit sur la sincérité de nos débats. Mais je m'interroge aussi sur la sincérité du ministre. Oui parce que le décret portant convocation sur le projet de loi signée par madame, la Première ministre, le 23 janvier 2023 et signé également par vous d'ailleurs, Monsieur le Ministre Dussopt mentionne le présent projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État sera soumis à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie que jeune sénateur je suis coupable de beaucoup de légèreté, mais je pense qu'il y a de la légèreté dans la façon dont on mène ce débat et qu'il y a un problème de sincérité réelle qui devrait exiger que sur tous les bancs de cette assemblée. On demande que cet avis ne soient transmis puisqu'il y a. Merci. Madame là. Présidente Rossignol pour un rappel au règlement. Dans l'article 33. Madame la présidente. En fait je vais vous demander une suspension de séance de 10 minutes pour 2 raisons, la première c'est parce que nous avons découvert effectivement une interview de Monsieur le Ministre, qui porte exactement sur les sujets que nous évoquons depuis jeudi et nous voudrions prendre le temps de lire cette interview parce que le plus souvent, les réponses que nous n'avons pas ici, on finit par les trouver dans le journal. Donc ça pourrait peut-être nous aider à accélérer les débats que de lire l'interview de Monsieur le Ministre. Et puis par ailleurs il faut quand même clarifier cette affaire Davy de notre que rendu public pas rendu public existe, il existe pas, c'est un 2ème sujet on comme je suis très économe de notre temps. Je propose qu'on traite dans la même. Suspension de séance soyez sont reconnaissants, chers collègues. Et donc, madame la présidente, je vous demande une suspension de séance de 10 minutes puisqu'il vous revient de nous l'accorder, ou pas, mais croyez-moi, nos collègues aussi seront probablement intéressés de prendre le temps de lire l'interview du ministre puisque nous plus que vous puisque le ministre-dit dans certains cette interviewe que cette réforme est de gauche, vous comprendrez bien que ça nous interpelle et nous avons besoin avec nos collègues des 2 autres groupes de gauche, de nous réunir pour vraiment expertiser cette affirmation et vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mensonge. Bon alors écoutez, moi je vais terminer. Les explications de vote et les votes sur sur les amendements, quant à. Étudier ou rue ou lire ses interviews où ces textes. Je pense que on peut le faire dans la nuit et demain matin vous pourrez redemande. Vous pourrez redemander Au président de de séance pourrait ainsi interrogé. Je, je ne suis pas sérieuse, je ne suis pas sérieux je le sais. Monsieur, ce n'est pas grave. Donc je décide et donc je vais faire ça n'est pas grave. Donc je vais mettre aux voix donc l'amendement 4019 avis défavorable de la commission du. Gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient pas adopté la on l'enquête 1100. Même avis même vote. Le 4025, même avis même vote. Je écoutez je, je ne sais pas ce que vous dites.

je vais mettre aux voix l'amendement 4106, ce qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Non. Adopté le 2746 qui est pour. Ah des explications de vote. Moi je veux bien, il y a pas de souci hein. Je ne vois pas de main levée. Non bah alors donc. Écoutez, moi j'ai mis en fait s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, qui représente la le groupe socialiste. Vous levez la main et vous me dites si vous êtes dans des scrutins publics etc. Plutôt que de m'empêcher de mettre aux voix sincèrement et de respecter un petit peu même la présidente Rossignol. Vous êtes des fois ma place, donc vous devez comprendre quand même.

Il y a pas de souci Madame Rossignol. Alors on en est aux 2746 on a on a une demande de. Non non non ben en plus il y a pas les bons numéros donc écoutez moi je mets aux voix le 2746. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 2749 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté. S'il vous plaît. Je vous ai pas empêché de parler tout le temps. vous sollicitez depuis le depuis hier un document moi sincèrement moi j'ai entendu les explications du ministre qui vous la donner, plus d'une fois du rapporteur, président de l'Amex. Voilà donc maintenant vous demandez des suspensions pour aller lire des publications. Écoutez, sincèrement, faut être juste un petit peu sérieux par rapport au sujet. Voilà donc s'il vous plaît. Oui mais. Il y a pas de problème Monsieur Bourgi. Hein vous arrêtez de m'interpeller. Pour commencer. Deuxièmement les suspensions de séance. C'est le président qui les donne. Donc voilà c'est tout. Maintenant, je vous demande de reprendre un peu votre calme. Et nous allons passer à l'amendement 2107. Oui Madame Lienemann.

pas. Nous avons écouté avec attention les réponses du ministre. Je vous rappelle ce qui nous a raconté nous a dit. Nous a dit, dans le cas d'un PLFSS. Il n'y a pas d'avis du Conseil d'État. Il y a une note de synthèse. Il nous a par ailleurs expliqué que quand c'était le le que la consultation du gouvernement. Une déclaration orale de Monsieur Hollande aurait décidé que c'était pas publié. Dans les décrets. Qui hein qui présente à l'Assemblée et au Sénat. Le PLFSS. Et cette se présente le PLFSS rectificatif. Il est explicitement cités. Après avis du Conseil d'État. vous voyez bien qu'il s'agit d'un terme juridique qui n'est pas tombé du ciel. Donc on peut s'interroger. Et on demande au ministre. De nous dire exactement s'il y a un avis ou pas du Conseil d'État. Et pourquoi. S'il y a pas d'avis. Dans le document qui nous est transmis. Il est fait référence à un avis nous n'avons toujours pas madame la présidente de réponse sur ce point. Avez. Madame de La Gontrie. Je comprends madame la présidente, que parfois ce soit un petit peu délicat de mettre de l'ordre dans certaines interventions et je comprends la difficulté de votre tâche nous demandons des scrutins publics et il serait vraiment bien pour la paix de cette discussion qu'il puisse avoir lieu. C'est un rappel au règlement. Alors sauf que comme. Je n'ai pas eu la parole du coup je n'ai pas pu garder la page sur l'Arctique sur les rappels. Alors écoutez. Vous ne faites rien depuis deux jours, nous nous travaillons. Madame de La Gontrie. Madame de La Gontrie. Je vais juste donner une précision quand même hein parce que les scrutins publics il y a aucun souci, je le dis au président ici. En revanche, quand on m'envoie des scrutins publics sur des numéros d'amendements qui ne sont pas ceux dont on parle là moi j'y peux rien mais voilà j'ai mis aux voix, on est bien d'accord que c'était pas les, les bons numéros. Voilà je vous remercie. 60 et 72 alinéa 2. Mais si. Monsieur Lemoine. Oui, sur la base d'articles 42 et suivants du du règlement. Madame la présidente. Puisque ce sujet. De la vie ou de la note. A été évoqué à plusieurs reprises. Nous sommes ici. Il y a une majorité sénatoriale. Il y a des groupes minoritaires, il y a une opposition les uns et les autres ont été amenés. Au fur Au fur et à mesure des années à exercer parfois les responsabilités exécutives d'autrefois. Ce sont les autres et donc je crois que nous avons tout intérêt à garder. Comment dire. Les équilibres qui sont ceux de notre constitution. L'article 39 de la Constitution qui prévoit que. Une loi organique défini les documents qui accompagne un projet de loi et en l'occurrence cette loi organique qui était débattu dans cet hémicycle qui était adopté par le Parlement ne prévoit pas que les lois de finances ou les lois de financement de la Sécurité sociale. Voit. Les notes. Divulguées et donc non. C'est un avis dès lors que c'est un projet de loi ordinaire. C'est une note dès lors que c'est un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais ce qui est important, je m'en tiens aux textes fondamentaux qui régissent les pouvoirs publics en France et auquel nous sommes donc ici je crois sur tous les bancs attaché il l'article 39 de la Constitution qui prévoit une loi organique. Cette loi organique elle été adoptée cette loi organique. Elle ne prévoit pas que. Les notes. Soient divulgués dès lors que le Conseil d'État et dans sa fonction de conseiller juridique du gouvernement et c'est très important que le Parlement, respecte la prérogative de conseil juridique du gouvernement, faute de quoi, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, c'est que le gouvernement, il demandera un avis qui sera un avis of il ne demandera plus des avis. En tant que telle au Conseil d'État et donc c'est très important, je crois que nous gardions ça en tête parce que encore une fois ici. La majorité d'un jour elle peut te la minorité du lendemain et vice-versa et donc ayons en tête l'article 39 de la Constitution cette loi organique qui fixe les principes et qui prévoit que cette note. Elle n'est pas divulgué. Mais par ailleurs. le président de l'la. A dévoilé un certain nombre d'éléments qui nous permettent, je crois, poursuivent l'examen du débat et des articles c'est ce à quoi j'appelle désormais. Merci. Alain. C'est un passé à l'amendement 2107. Vous avez déjà fait un rappel au règlement. Madame de La Gontrie. Bon allez une minute. Second point et de ce point de vue, je pense qu'il est utile. C'est sur le 24 alinéa 2. De dire que ce qui a été. Jean-Baptiste Lemoyne, on peut le comprendre. Mais ça n'est pas adapté. Parce que ce qui est en question, ici, ce n'est pas de savoir si la publicité est obligatoire. La question, il est de savoir, elle est de savoir si le ministre n'a pas dit la vérité.

Vous ne l'aurait pas car il n'a pas d'obligation publicité on aurait pu apprécier polémiquer contesté ce n'est pas ce qui nous a été dit, il nous a été dit, il n'y a pas d'avis. Il a simplement une note. Or, Marie-Noëlle Lienemann, vous la luge vous suggère d'aller sur le site de l'Assemblée nationale et vous verrez le fac-similé du projet tel qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale et qui dit expressément que le texte a été adopté en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Donc le point qui est aujourd'hui soulevée madame la présidente, c'est de savoir pourquoi le ministre nous a dit autre chose que la vérité qui sauf à nous dire que ce qui est écrit dans le document du du de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui suffit Monsieur le Ministre. Madame de La Gontrie sincère. Interpellé par le ministre. Non mais vous l'avez hein interpellé est ce que vous avez dit, n'est pas très respectueux

S'il vous plaît. Je vais donner la. Parole au président Gontard pour un rappel au règlement je donnerai ensuite la parole à monsieur le rapporteur. Savary et ensuite à Monsieur le Ministre et ensuite je donnerai une suspension de séance de cinq minutes, voilà. Si le président Gontard.

quand même, je veux dire on nous a expliqué, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, je sais plus le temps passe, le temps passe vite on a demandé très clairement. L'avis du Conseil d'État. On a demandé à plusieurs reprises on a eu une intervention du ministre qui nous a expliqué qu'il a expliqué ça de manière très claire d'ailleurs hein, que ce n'était pas un avis, il nous a expliqué pourquoi. Ce n'était pas un avis que c'était une note et pourquoi on ne pouvait pas obtenir cette note on apprend et on regarde très clairement que bah si c'est un avis, donc je pense qu'à un moment donné il y a une vraie question de sincérité et derrière tout ça, je veux dire quand on voit ce texte. On a parlé de l'Assemblée nationale. Mais le nombre je dirais de de contrevérités en tout cas qu'il peut y avoir de ce texte les approximations qu'il peut y avoir, je pense que ça commence un petit peu à bien faire, on est a priori sur un texte sérieux, qui concerne quand même la vie des gens et je pense qu'à un moment donné, on est en droit d'avoir de la vérité, d'avoir une réponse claire et c'est pas la question d'attaquer quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est d'avoir des réponses claires. On est ici pour pour débattre. accordez vous voulez vous souhaitez nous accorder une suspension de séance. Je voulais vous le demander, ce que je pense qu'après les interventions du je pense qu'on aura besoin de cette interruption de séance à la fois pour que les débats puissent bien se passer et puis qu'on puisse discuter tous ensemble. Merci. Merci. Alors je donne la parole à monsieur le rapporteur. Savary. Merci madame la présidente. Jusqu'à présent nos débats s'était bien passée. Relativement bien passé. Parce que à un moment. Vous avez parlé d'un silence mensonger. Qui est limite dans l'expression que nous devons avoir ça n'amène rien au débat. Ceux qui nous regardent. Je pense. Émettent un avis plutôt défavorable par rapport à la qualité de nos débats, c'est pas acceptable. D'autant plus que on voit bien que cette réforme touche nombre de personnes. Maintenant, madame de La Gontrie. Vous avez dit qu'on faisait rien. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. De façon générale, nous travaillons toujours ses textes on le travaille depuis 4 ans, 5 ans, ce texte. Ça vous a échappé. Vous voyez-vous ça montre bien, ça montre bien, ça montre bien que vous préférez les effets de tribune à l'efficacité du travail. Maintenant quant à la transparence. À propos de cette note. Une note c'est une note. Mais vous le savez bien.

N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour lire le monde pour ceux qui ne l'ont pas lu tout et explique cite ment décrit dans ce journal et vous le servez pertinemment et il n'y a rien de plus en plus, il y a des membres du de la makes qui peuvent venir me voir et ils auront. Les explications autour de cette note dans la plus grande confidentialité qui est la même confidentialité. Que le secret fiscal que connaissent bien le président Reynal ou le président et blé. Alors qu'on ne n'arrêtent de nous donner des leçons. Merci. des leçons. Merci. Merci madame la présidence, c'était simplement pour confirmer hein. Mesdames et messieurs les sénateurs que le document que le Conseil d'État a transmis au gouvernement pour donner son appréciation sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif est une note. Qui a été approuvé par le Conseil d'État dans sa séance du 19 janvier. Une fois j'ai dit cela. Est remise en cause de la sincérité, l'honnêteté. J'avais cru comprendre que je n'étais pas l'Assemblée nationale. Mais monsieur le rapporteur. La rappeler avec. Très bonne décision. Merci Monsieur le Ministre. Alors je vais suspendre la séance pour cinq minutes séance est suspendue.

je souhaite que nos débats, concerts, la sérénité qui fait la marque de fabrique de notre assemblée et contribue à la bonne image ne nos travaux alors je n'hésiterai pas enfin de maintenir la sérénité de nos débats à faire usage des prérogatives que le règlement confère à la présidence de séance. Mais ce rappel ayant été fille nous reprenons le cours normal de la discussion. Monsieur Lurel. Merci madame le président et j'espère que vous croirez qu'il ne s'agit pas. De. Porter atteinte à la sérénité de nos débats. Mais c'est vrai lorsqu'il y a. Incompréhension, il faut aller au bout d'une explication. On a entendu et je crois que chacun ici est de bonne foi, moi j'ai consulté la loi organique suggéré par note. Collègues. Celle de du 15 avril 2009 sur la présentation des textes pas de notes. On ne dit pas. On parle d'impact. Pour les projets de loi et on dit que à l'article 8 de cette loi organique à l'article 11 de cette loi organique que ça ne s'applique pas aux lois de finances aux lois de financement à la révision constitutionnelle aux traités internationaux de l'article 53. Mais à aucun moment on ne parle d'avis cet avis doit être donnée, c'est les études d'impact qui ne s'applique pas mais la vie doit être communiqué. Ensuite on a inventé la notion de notes. Et voilà je suis un peu étonné, j'ai cherché ou est-ce que ça existe. Je ne l'ai pas trouvé. S. troubler la sérénité de nos débats, que de demander une clarification. C'est quoi la note de synthèse, elle vient d'où elle sort d'où elle figure dans quel texte. La note de synthèse moi ici dans cette loi organique d'ailleurs très largement censurée par le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas donc j'aimerais avoir cet avis. Merci. Alors on va passer à l'amendement 2107 présenté par Madame la rapporteure pour la commission. Oui c'est un amendement correctionnel madame la présidente. Tu y as monsieur le vous rappelons favorable. Je vais donc on voit cet amendement. Donc de la commission et avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contraint qui s'abstient. Il est donc adopté. J'ai passer au vote sur l'article 1er. Madame Lienemann. On a eu une discussion approfondie. Sur la remise en cause des régimes spéciaux. Mais il est bien apparu aux uns et aux autres. Que le coeur de ses remises en cause. Concernés à la fois les salariés de la RATP. Et ceux des industries électriques et gazières. Or ce n'est pas une mince affaire. De remettre en cause. Ce que notre collègue. Pierre Laurent a appelé le pacte. Entre les salariés de ce secteur. De ses piliers de service public. Et l'impérative nécessité qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. A consolidé. Et ses services publics et de relever les défis tant des transports que de la question énergétique. Il y a un parallélisme. Entre la remise en cause. Par la marchandisation la financiarisation de ces régies de ses services publics. Et le décrire tricotage du modèle social des salariés de ce secteur. Vous êtes dans un mécanisme où ce qui a fait la force. Les fondamentaux de notre République. Qui sont aujourd'hui considérablement affaibli par les politiques néolibérales vont encore subir un mauvais coup à un moment il me faudrait relever les défis. La 2ème chose c'est le rapport à la pénibilité. Car vous vous attaquez à des métiers des emplois des salariés qui ont une vie difficile au travail. Qui ont des contraintes qui ont de la pénibilité. Or tous les mécanismes généraux de pénibilité que vous mettez en place sont jamais qu'au bout du compte l'ultime réparations potentielles de la dégradation liée à leur travail, alors que ce statut conclure leur garantissait au contraire une vision plus préventive et protectrice. Oui merci madame la présidente sur cet article premier je voudrais repréciser au terme de son examen quelques points. Je voudrais rappeler qu'il y a quand même 500.000 cotisants tous régimes spéciaux confondus. À mettre en rapport au 28 millions de cotisants d'autres régimes, la suppression donc des régimes spéciaux de retraite et on l'a dit à plusieurs reprises un serpent de mer qui se nourrit des rockers et et des rancoeurs et qui se nourrit des ressentiments et ce n'est pas un hasard si la suppression de certains de ces régimes et des y'discuter dès l'article 1er de ce projet de loi. Toutefois, si nous pensons que le gouvernement joue un jeu dangereux en opposant les Français entre eux, il n'en demeure pas moins que la mobilisation des mondes qu'aujourd'hui cette stratégie ne fonctionnement ne fonctionne pas et je le redis, nous en aurons encore la démonstration sans aucun doute mardi prochain. Nous n'avons eu de cesse de dire les raisons pour lesquelles vous souhaitez supprimer ces régimes spéciaux mais mais pourtant. Il nous reste encore un certain nombre d'interrogations pour lesquels nous n'avons pas eu de, de réponse une suppression à la carte au nom de l'équité. Mais pourquoi ne pas réformer tous les régimes spéciaux, pourquoi en préserver certains et pas d'autres. Où est la justice lorsque vous supprimez de manière arbitraire cinq régimes spéciaux sur 17 ans maintenant donc douce et Charles de Courson qui disait ça à l'Assemblée nationale, toujours au nom de l'équité entre tous les Français, le gouvernement veut mettre fin aux régimes spéciaux supprimer des acquis des uns ferait donc le bonheur des autres. Qu'en est-il des retraites chapeau et autre parachutes dorés. Dans ces cas-là, parce que les régimes spéciaux sont déficitaires. Cela n'est pas vrai. Plusieurs d'entre eux sont, nous l'avons démontré pourtant excédentaire et pourquoi vouloir à tout prix. Mais tout le monde, aux mêmes conditions minimales prévues par le droit du travail, en rejetant les conventions collectives qui améliorent. L'ordinaire donc sincèrement, nous n'avons pas eu de réponse à toutes ces questions et c'est une des raisons supplémentaires pour lesquels nous voterons contre cet article 1er. Merci madame Cohen. Oui merci madame la présidente, en fait. Le fin mot de de cette suppression des des régimes spéciaux. C'est que il faut tirer tout le monde vers le bas et faire travailler plus. Et pour plus longtemps et c'est l'horizon qui est proposé par ce gouvernement et soutenu par la droite et on l'a bien vu puisque le le rapporteur nous a dit que ça faisait 5 ans que vous travaillez sur ce projet de loi, donc on comprend maintenant la connivence qui existe entre le gouvernement et le vent de de la droite mais la question qui est posée, quand même, c'est est-ce qu'on peut vraiment travailler jusqu'à 64 voire 67 ans, quand on sait que le taux d'emploi des seniors n'est que de 56% en 2021 selon la Darès faut-il vous rappeler que lors du précédent allongement de l'âge légal de la retraite à 62 ans le taux de chômage des plus de 55 ans a bondi de 23% en 2011. Un nouveau recul de ce seuil pourrait donc avoir pour conséquence d'accroître encore le chômage des seniors. Comme le souligne l'économiste Michaël Zemmour à partir des travaux de l'adresse et de la Darès le coût social du décalage de l'âge minimum de la retraite à 64 ans, ce sera une hausse de l'ordre de 100.000 du du nombre d'allocataires de minima sociaux, 120.000 pour les pensionnés d'invalidité supplémentaires auxquels il faudrait ajouter une hausse du nombre de chômeurs indemnisés et de personnes sans emploi mais en mais n'ayant droit à aucune prestation spécifique le tout représenterait environ 300.000 personnes de plus maintenus dans la précarité entre emploi et retraite. Enfin vous répéter à l'envi que les régimes spéciaux coûtent 1,8 milliards aux contribuables. Mais alors que dire de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a coûté près de 4 milliards aux contribuables du CICE, près de 20 milliards de cotisations et les aides publiques aux entreprises sans aucune contrepartie, ni sociale ni environnementale, ce sont 200 donc ça fait beaucoup. Vous voyez pour de l'argent qui manquait. Voilà une note que je vous offrent sur un plateau. Merci madame Lubin. Maintenant que nous arrivons à l'issue de cet article de suppression des régimes spéciaux, moi la seule chose que j'ai envie de dire c'est ça lui et vous y serait arrivé si. Ce. Projet de loi venait à être voté ce que pour l'instant je ne souhaite pas Il y a des chances ou des risques qu'ils le soient selon le côté duquel on se, on se pose. Vous y serez arrivé j'allais dire que cette espèce de serpent de mer. Cette espèce de de souhait que vous aviez depuis. Depuis très longtemps. Il aura suffi. D'un petit projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale puisque je vous rappelle qu'on est toujours là dessus, il aura suffi de de de ça de ce de ce petit texte dans le Dont vous profitez pour repousser l'âge de la retraite de 2 ans, il aura suffi de ça pour que. Vous arriviez. À mettre fin. À des régimes de retraite historique et protecteur. Concernant des pans extrêmement important de notre économie mais aussi. D'une autre comment dire de notre richesse sociale, j'ai envie de dire. La RATP le régime des gaziers. Franchement si vous y arriver. J'aurais presque envie de dire chapeau les artistes. Parce que là où tous vos prédécesseurs auront échoué. Vous finalement. En peu de temps. Vous y serez parvenu alors j'espère que notamment tous ceux qui sont concernés feront entendre suffisamment leur voix, encore plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant dans les jours qui viennent et nous nous faisons entendre la nôtre dans cette assemblée. Mais. Franchement je je ne sais pas si vous vous rendez compte. De quoi vous serez comptable à la fin. Merci monsieur Chantrel. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, je vous ai interpellé tout à l'heure poliment. Concernant votre entrevue. Dans un journal qui paraît demain. Vous vous dites que la réforme ne fait aucun perdant. Je constate que j'avais donné des points précis. Vous n'avez répondu sur aucun point. C'est normal, je pense que ça vous très très très très mal à l'aise puisque. Elle ne fait que des perdants. Y compris. Ceux qui sont concernés par cet article 1. Concernant les, les régimes spéciaux. La vérité que vous refusez de reconnaître quoi quand elle vous dérange c'est que. On l'a répété tout au long de. Depuis le début de la discussion c'est que vous vous servez des retraites. Pour rembourser des baisses d'impôts qui favorise les plus riches. C'est ça le but. De votre réforme. Elle est injuste à la inéquitable aggravera la situation des femmes, des Français qui ont une carrière hachée ou une carrière longue et de ceux qui exercent les métiers les plus difficiles et qui sont concernés également. Par cet article le premier justement. Vous maquiller la vérité. À longueur de journée pour faire passer la pilule, mais celle-ci devient de plus en plus indigeste. C'est pour ça que nos compatriotes. Sont de plus en plus nombreux dans la rue. Pour manifester contre ces réformes et nous serons à leurs côtés. Pendant les pauses. Mardi prochain. Bien évidemment, pour que vous retiriez cette réforme. Injuste. Ça es forme allez aussi brutale qu'impopulaire. Personne ne peut accepter de perdre 2 ans de retraite bien méritée. Quand les dividendes des entreprises du CAC 40 explosent sans subir aucune surtaxation donc écouté les Françaises et les Français qui sont massivement contre cette réforme est retiré là. Merci monsieur le questeur bah. Merci madame la présidente. Nous arrivons à un moment important de ce débat avec le vote sur l'article. 1er. Et je voudrais tenter un exercice qui ne me paraît pas impossible. Faire ressortir ce qu'il y a eu de positif. Dans ce débat. D'abord j'en retiendrai que sur cette question qui n'est pas celle de la suppression. Des régimes spéciaux mais seulement celle de leur fermeture. À compter du 31 août prochain. Il y a. Non pas. Une approbation générale. Mais au moins une acceptation. J'en veux pour preuve d'admirables amendements je citerai. Le 3045, signé par monsieur Kanner. Et le 3913. De la présidente Assassi qui l'un et l'autre reporte cette fermeture des régimes spéciaux, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on ne peut plus avoir de nouveaux entrants dans ces régimes. À l'échéance du 31 décembre 2027 et non plus du 31 août 2023. C'est dire chers collègue qu'il y a, comme l'a dit Madame de La Gontrie tout à l'heure un chemin qui s'est ouvert aujourd'hui. Et Monsieur Didier Marie. Et monsieur Didier Qu'on s'achemine vers une forme de compromis malheureusement une journée n'aura pas suffi pour qu'on s'entende sur cette date mais à tout le moins, soyons fiers d'avoir fait émerger une forme de consensus sur le principe de la fermeture des régimes spéciaux quant à leur disparition. Ah l'a été votée en 2010. Je n'ai pas le souvenir que quand la gauche a été au pouvoir, elle en est remis en cause le principe, nous en discuterons après l'article 7 sur le fondement de l'excellent amendement du président Retailleau. Merci madame monsieur. oui merci madame la présidente. Cette. Proposition. Elle est injuste et injustifiée, je l'ai souvent dit. Elle est injuste envers les femmes particulièrement envers les jeunes pour certains territoires parce qu'il y a un taux de chômage important et quand on voit ce qui est proposé, hé bien c'est vraiment dommage que le gouvernement. La rapporteure et tous les autres n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer concernant. Les régimes concernant les régimes et le d'électricité et de gaz mais surtout l'électricité. Il y a une tendance à l'externalisation. La Première ministre, madame Borne avait évoqué et avait demandé la sobriété énergétique, il y a quelques mois, la souveraineté et pourtant la résultante de notre façon d'anticiper et voir s'attaquer au modèle de retraite de ces filières très utile pour le développement économique et géostratégique c'est c'est une erreur très importante et surtout très grave. Vous allez tuer l'attractivité vers les métiers. Importants pour notre développement limité au niveau systémique à terme l'aménagement du territoire également parce que l'électricité c'est important pour l'développer l'aménagement. Cela va également porter sur les effectifs et si les prévisions des emplois et des compétences parce que personne ne voudra rentrer de ce système. J'appelle à la raison. Nous devons protéger ses systèmes. Pour notre propre devenir. Externaliser. C'est une erreur très grave qui sera irréversible systématiquement. Oui merci madame, la la présidente. C'est vrai que sur cet, cet article 1 qui n'est, qui est loin d'être anodin sur le revenir sur ces, sur ces régimes spéciaux. Je pense qu'il y a plusieurs aspects, déjà il y a évidemment un, un jeu dangereux à la fois sur sur le clivage qu'on n'essaie de faire monter entre les Français les uns contre les autres et je pense qu'on est vraiment pas dans une période où on a besoin de ça. D'opposer déposer les les les Français à travers, à travers À travers leurs avantages, mais qui ne sont pas des avantages n'importe quels avantages sont les avantages qui ont été qui ont été acquis. Et puis surtout, ces régimes spéciaux. Ben ils ont une vraie est un vrai intérêt notamment sur l'attractivité de ces métiers et, pour la plupart de ces métiers. On l'a vu pour. Pour les et les Christian l'a vu pour la RATP, ce sont des métiers évidemment. Essentiel et dont on a un besoin essentiel. Donc je pense que ça serait une grave erreur de revenir sur ces aspects-là et puis. Je pense qu'il y a un problème de à la fois de cohérence et et d'analyse parce que je ne vois pas comment on peut intervenir globalement à la fois sur la RATP électriciens le 16. Les clercs de notaires avec des régimes qui sont tous totalement différent et donc ça me paraît difficile de pouvoir délibérer sur cette cette question là. Et puis en même temps on n'a aucune aucune analyse financière. J'en prends pour exemple la réforme du CESE je crois de 2015. Sur lequel il y a eu des grosses modifications on a aucune évaluation. Il me semble avoir vu aucune à la fois qu'une évolution financière qui une évolution sur la trajectoire de ce de de ce régime. Donc comment on pourrait vouloir le modifier sans savoir exactement où il en est et puis derrière tout ça et notamment derrière sur le régime à la fois de la RATP sur le régime des électriciens et des gaziers et ben on le sait très bien que c'est revenir sur un statut et un statut eux important sur à la fois la dépendance des des fonctionnaires. Donc pour toutes ces raisons évidemment s'opposera sur cet article 1er. Merci madame la présidente Rossignol. Madame la présidente. D'abord une petite remarque, je propose qu'on observe ensemble la vertu apaisante d'une petite suspension de séance de cinq minutes. Mieux qu'une tasse de passiflore. et nous nous retrouvons là tous dans un débat courtois comme nous aimons en avoir pour autant que courtois que soit le débat il ne doit pas dissimuler nos divergences profondes. J'admire l'effort fait par le questeur bah qui décidément s'impose. Également dans cet hémicycle comme un homme capable de bâtir des. Compromis. Mais pour autant je dois lui dire que en ce qui concerne les amendements qui a cité. Je ne lui ferai pas l'insulte de ne pas savoir ce qu'un amendement de repli mais comme vous avez remarqué probablement aussi vos téléphones portables que beaucoup de gens nous regardent, nous recevons tous de nombreux SMS commentant nos interventions les uns et les autres et la qualité de nos débats. Alors pour ceux qui nous regardent, je vais quand même préciser que ces amendements qui effectivement. Changer la date d'application de l'extinction des régimes spéciaux et ce qu'on appelle dans notre jargon des amendements de repli qui vise effectivement à essayer d'atténuer un peu, une disposition que nous critiquant. Ceci étant dit, pourquoi nous allons voter contre cet article hein parce qu'il concentre il est emblématique de l'idéologie de ce projet de loi. Son idéologie. En fait, elle consiste à ne pas prendre en compte les corps intermédiaires et changer le régime du CESE sans leur demander leur avis. Elle consiste à s'attaquer principalement au régime des gaziers des électriciens et c'est bizarre parce que c'est toujours les mêmes gaziers les mêmes électricien tous ces salariés qui sont effectivement structuré par une histoire sociale importante qui sont montrés du doigt comme étant ceux qui résistent le mieux aux offensives libérales des gouvernements et eux aussi, vous voulez les attaquer donc les corps intermédiaires, les pôles de résistance du ça n'est plus avancée du salariat. Tout est concentré dans cet article hein pour pouvoir ensuite déboucher sur l'article. Ce cette qui est la grande offensive de votre projet. Le report de l'âge de la retraite. Merci, Monsieur le comte. La présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues d'une réforme. Nous l'avons déjà dit hier qui est d'abord là pour masquer. Une mauvaise gestion, essayer de récupérer quelques milliards. Perdus par ailleurs parce que. Non pris là où il y a des profits. Parce que des cotisations ont été abaissées parce que des salaires. Au lieu d'être augmenté. Hé bien. On multiplie les primes. Qui n'abonde pas ensuite les caisses de la Sécurité sociale. Voilà alors puisque il manque de l'argent, c'est les plus faibles derrière qui qui paieront. Et voilà la première étape. On choisit certains régimes. Spéciaux de la sécurité sociale. Alors certains qui fonctionne bien. D'autres. Qui prennent en compte la pénibilité, la dangerosité. Je pense en particulier à celui des industries électriques et et gazières qui. Sait prendre en compte un certain nombre de de points de manière bien différente que le régime général en particulier depuis l'ordonnance de 2017 qui a supprimé un certain nombre de critères de de de pénibilité. Alors voilà. Par cet article. On supprime l'entrée dans des régimes plus protecteur ou des régimes qui fonctionne le droit à entrer à un certain nombre de personnes alors que. Sur un certain nombre et en particulier sur dans le domaine de l'énergie, nous avons des difficultés de recrutement, nous avons besoin de de renforcer notre service public. De l'énergie et la suppression de de de de ce régime ne sera pas une une bonne idée en opposant les uns avec les autres en montrant du droit, ce qui vont être. Qui ne pourront pas bénéficier de ces régimes spéciaux parce qu'on leur a dit que finalement leurs aînés étaient des privilégiés, on a monté les uns contre les autres, ce n'est pas de cette manière-là qu'on construit la cohésion du pays ce n'est pas de cette manière-là qu'on construit la confiance et c'est parce que nous souhaitons si cohésion sociale dans le pays. Sur le compte ne l'ont pas monsieur le comte c'est bon maintenant on va laisser la parole à Madame Ferré. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Je veux rappeler tout d'abord, c'est une évidence. Ce premier article de la réforme, hé bien c'est tout tout simplement supprimer les régimes spéciaux. Alors voilà un symbole très fort, je rappelle que ces régimes spéciaux ont été instaurées au moment de la création du régime général de la Sécurité sociale en 1945 cela en reconnaissance de contraintes professionnelles qu'il s'agisse d'horaires décalés, travail de nuit, de conditions de travail spécifique à certaines professions. Maître remettre pardon en cause ces régimes spéciaux oh sous prétexte d'équité ou de supposés universalité est véritablement une diversion de votre part pour faire oublier que cette réforme votre réforme hé bien c'est tout simplement 2 ans de plus pour tous. Nous n'en voulons pas. En fait c'est une fois de plus pour vous l'occasion de diviser les Français, entre ceux qui seraient privilégiée et les autres mais. Privilégié quand on vit au quotidien des conditions de travail des, de la pénibilité réel qui est constaté. Mais il est vrai que cette notion de pénibilité. Vous êtes étrangère puisque maintenant on parle d'usure professionnelle puisqu'en 2017, vous n'avez pas hésité à supprimer 4 critères de pénibilité sur 10. Alors vous ne reconnaissait pas ainsi cette pénibilité dans de nombreux métiers, vous remettez en cause véritablement le contrat social des salariés avec leur entreprise vous décider unilatéralement, sans concertation avec les organisations de ces fermetures ou de de Cesare de régimes spéciaux vous pénaliser des secteurs d'activités stratégiques pour notre pays. Ça a été évoqué. Alors comment rendre aussi plus attractif ces secteurs d'activités qui rencontrent déjà des difficultés à recruter. Enfin, je voudrais terminer parce que vous nous avez conseillé les uns et les autres, de lire la presse, effectivement ce soir, le JDD a publié un sondage qui dit que seulement 32% des Français se disent favorables à votre réforme, alors il est encore temps. Réagissez. Mais elle rire quoi qui reste cet article Merci madame la présidente. Donc cet article 1 prévoit la suppression des régimes spéciaux de retraite pour les personnes nouvellement recrutés à compter du 1er septembre 2023. Il va de Pair avec l'article 7, que nous examinerons dans quelques jours puisque vous souhaitez appliquer aux régimes spéciaux les mêmes dispositions et à les intégrer dans le régime général. Le gouvernement considère que l'existence de ces régimes spéciaux n'est plus justifié et serait inéquitable inéquitable pour notre modèle social. Nous avons une différence d'appréciation et c'est normal puisque vous êtes unis à droite dans ces bancs sur ces bancs et nous sommes unis à gauche. Loin d'être des privilèges, comme vous le prétendez, ces régimes spéciaux ont été créés pour mieux compenser la pénibilité des métiers qui sont exercés dans les fêtes, les régimes spéciaux ne concerne pas l'ensemble des salariés du secteur. Mais ceux qui ont des conditions de travail les plus dures et des des suggestions spéciales donc non seulement à son arrivée au pouvoir en 2017, le gouvernement a supprimé la reconnaissance des quatre critères de pénibilité mais vous supprimez tous de la compensation de la pénibilité des métiers existantes, par le biais des régimes spéciaux. Vous choisissez de supprimer 5 régimes. Spécial cinq régimes spéciaux, la RATP, les industries électriques et gazières. Celui des clercs de notaire des membres du CESE, de la Banque de France. Vos arguments ne nous ont pas convaincus, et nous, nous nous ne pourrons pas voter cet article 1 qui est une règle une régression. Pas de dialogue social. Pas d'évaluation. Financière. Une réforme qui fera des perdants et des perdants 5 fois des perdants. Pour ces cinq régimes spéciaux donc nous voterons contre cet article hein. Merci madame Préville. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord je souhaiterais intervenir pour parler de 2 sujets majeurs dans notre actualité qui concerne à la fois les transports et énergie. Ce sont des sujets très importants dans notre société et très. Singulièrement les régimes spéciaux qui sont attachés à ces 2 grandes familles de salariés sont attaqués. C'est oublier le bénéfice dont nous avons largement profité. Nous avons un cruel besoin de services publics de transport solide et efficace pour lutter contre les gaz à effet de serre, ça c'est la première chose 2ème chose. Avez-vous mesuré les conséquences de la fermeture du régime spécial des électriciens et des gaziers toute la filière de l'énergie va être fragilisé et quel avenir énergétique. La France peut à la voir dans ces conditions. Pensez-vous. Faire au sujet et au, au vu du mur des investissements qu'il nous faudra faire. Auquel il ne faudra faire face, de pouvoir faire au rabais et à moindre coût, comme si construire des centrales nucléaires, des installations de stations électriques par pompage n'étaient pas des enjeux industriels conséquent. Nous avons par le passé. Connu de belles réussites parce que nous avions des salariés protégés des salariés reconnus bien dans leur travail et fiers de leur travail. Ce fut. Ce fut certainement le gage de réussite que nous avons connu et nous prenons ainsi de nombreux risques très inquiétant et je le rajoute. La suppression de l'IRSN, qui est vous savez, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un institut indépendant de recherche et d'expertise finalement qu'est-ce qui a failli dans tout cela. apparemment il n'y avait pas de raison. À vrai dire. Principalement, on peut mettre en cause la sous-traitance et la fin de cet institut qui sont très préoccupante. Donc voilà c'est pour cela et je terminerai sur les et la fin de ce régime parce que suite à l'intervention. Merci maman. Merci monsieur Cabanel. Oui merci madame la présidente. Monsieur le. Le ministre. L'article 1 vise à supprimer certains régimes spéciaux. J'ai bien hein. Entendu tous les arguments que vous avez donné les uns et les autres. Parfois des arguments très. Et très similaire d'ailleurs. Et vous avez parlé de pénibilité d'injustice et la pénibilité. Je vous rejouer sur sur ce mot mais je pense qu'il y a un article, l'article 9 sur lequel on pourra évidemment parler de de pénibilité. Certaines d'entre vous ont avancé comme argument que. Il était donc difficile de recruter et si on voulait donc pouvoir recruter il fallait garder ces régimes spéciaux. Je pense pas que ça soit le problème du recrutement qui touche exclusivement les régimes spéciaux. En agriculture, en manque de recrutement dans l'Éducation nationale au manque de recrutement dans la santé, on manque de recrutement et je m'arrêterai là. Donc moi je suis dans une logique de de de simplification d'harmonisation. Et de de solidarité que les régimes spéciaux soit autonome ou pas.

Parce que c'est un travail suffisamment pénible mais je je moi je crois que on pourra parler effectivement de pénibilité à l'article 9 et c'est pour cela qu'à mon âme et conscience, je voterai pour cet article. Merci monsieur Redon Arazi. madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après une journée de débats j'allais dire mais mais non pas de débat parce qu'il y en a pas. Donc une journée d'explication des amendements déposés par cette partie de l'hémicycle. Nous avons nous prononcer sur cet article vous avez placé en premier l'article sur la gym spéciaux. C'est sans doute pas. Un hasard vous présupposé une adhésion de l'opinion à cette mesure. Vous êtes sans doute un peu trop optimiste. Nous sommes depuis le début de de de nos échanges. Et croyez-vous que que les Français et les Françaises qui sont particulièrement inquiets quant à leur budget énergie et qui nous regardent et qui il y a quelques semaines. Subissait les alertes de l'exécutif sur les risques de coupures de l'approvisionnement électrique sont prêts à tenir les personnels des industries électriques et gazières comme responsable de la situation qu'ils connaissent en raison de leur système de retraite. Je peux vous dire, c'est non. Et croyez-vous aussi qu'il considère. Que les agents de la RATP et le régime de retraite sont responsables de la prime de transport, pas plus. Eh bien nous nous avons la faiblesse d'écouter ceux qui seront dans la rue mardi prochain et même ceux qui ont d'ores et déjà commencé. La contestation et nous ne voterons pas cet article. Merci madame la présidente. Cet article hein. C'est donc la remise en cause des régimes spéciaux. C'est-à-dire la la remise en cause d'un pacte social et surtout la remise en cause des services publics en particulier, cela a été dit par mes collègues. On a parlé beaucoup ce soir de humilité mais vous vous ne tenez pas compte et vous avez même dès 2017, supprimer quatre critères de pénibilité. Ceux-là même qui provoque le plus de maladies professionnelles et côtes donc le plus cher à notre sécurité sociale. Si cet article. Venait à être votée. Je crains malheureusement que ce soit le cas, vous aurez gagné comme l'a dit mon collègue Monique Lubin vous aurez tué les régimes historiques et tout cela dans un seul but bien réel, lui lui qui le diminuer les déficits publics parce que oui, vous avez mis à mal par votre politique de cadeaux fiscaux et d'exonérations de cotiser social toutes nos finances publiques.

ils sont intelligents ils sont informés. Et il se pose la question du pourquoi. Quelle est la philosophie qui sous-tend cette urgence à traiter ce sujet globale des retraites et plus précisément des régimes spéciaux. Maintenant. La justice va mal. Les prisons sont encombrés. Les gardiens font défaut. La santé et les hôpitaux. Il ne se passe pas une journée sans qu'on cite le drame dans lequel et notre service public en matière de santé, la sécurité ne va pas bien. Les recrutements sont difficiles. Les salaires sont bas. Et plutôt que de se préoccuper en chambre de savoir comment on peut corriger. Tous ces problèmes, on remet une couche en disant on vous supprime les régimes spéciaux, on vous supprime et on vous met 2 années de plus de travail et. On, on vous demande d'accepter ça comme si de rien n'était. Et bien non. Malgré toutes les explications qui sont données. Les Français n'accepte pas tout simplement parce qu'ils savent, c'est que derrière la philosophie qui sous-tend tout cela c'est le la mise à bas du service public pour tranquillement glisser vers les services privés qui aux yeux de la majorité ici serait dans les temps futurs. Plus efficace plus productive et sans doute. Meilleur pour les rendements. Des des actionnaires parce que quand on parle de la valeur travail. qui remplit les esprits ici en disant la valeur travail de leur travail, moi je crois que c'est surtout la valeur des dividendes qui occupe les esprits de tous et de chacun et comment mieux rentabiliser les choses. Monsieur le Ministre, vous disiez hier. 17 milliards, c'est très important et, bien sûr mais.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voterai contre. Cet article Bien entendu, d'une régression sociale, mais surtout d'une offensive idéologique du gouvernement contre ces régimes spéciaux. En témoignent les déclarations du ministre du Travail, les régimes spéciaux sont devenues archaïques. La réalité des métiers évoluer. Faire cela, c'est avoir le courage que personne n'avait eu jusqu'alors. Je cite maintenant le ministre de l'économie c'est moi un problème financier que d'équité et enfin tout à l'heure. Monsieur Dussopt nous a indiqué qu'il y avait une rente dans les régimes spéciaux. Pourtant, ces régimes spéciaux on disait ont déjà connu de nombreuses réformes. Allongement des durées de cotisation baisse. Des taux de pension tous ont contribué à faire des efforts. Ces régimes spéciaux, nous l'avons déjà dit, c'est le fruit de nombreuses conquêtes sociales il nous sommes qu'aujourd'hui nous sommes revenus au temps des régressions sociales parce qu'il y a d'autres métiers qui sont également pénible on ne devrait plus reconnaître la pénibilité de ces régimes spéciaux. Non je ne crois pas, je ne crois pas que l'on doive tirer vers le bas l'ensemble mais plutôt aligner. Les pensions, les durées de cotisations. Sur les régimes spéciaux, il faut aller plutôt vers le haut que vers le bas, on a des problèmes de recrutement. En effet, dans de nombreux secteurs et les conditions de travail y sont pour quelque chose, je vous remercie. Merci monsieur dessus. Merci madame la la présidente. Mes chers collègues. Depuis la fin de cette soirée. On a basculé dans autre chose, on a un ministre qui fait la une. D'un quotidien demain en présentant cette réforme comme une réforme de gauche. On a un collègue questeur Monsieur bas qui nous dit qu'il y aurait un consensus entre les groupes de de cette assemblée et donc je me demande si je ne suis pas dans un univers parallèle. En réalité, en réalité, on a un ministre qui continue de jongler avec ses approximations ici comme à l'Assemblée a essayé de nous enfumer sur des détails. On a un questeur bah qui nous parle d'un consensus sur des amendements qu'il n'a lui-même pas voter ni son groupe conformément à leur stratégie de majorité silencieuse.

qui est de diviser en début de texte. Alors notre collègue nous l'a dit la pénibilité. On va, on va en parler au moment de l'article 9 mais d'abord il faut taper sur les régimes spéciaux mais pas n'importe quel régime pas n'importe quel régime la RATP et et l'énergie, la RATP, les transports en commun, l'énergie l'électrification de notre pays. Et donc là on voit bien qu'on a un gouvernement qui continue dans son déni des enjeux climatiques qui continue dans son déni de la situation sociale et donc dans un texte comptable. brutale une mesure brutale et injuste. Comme tout le reste du texte, il ne fait que des perdants. À commencer par les générations futures. Je vous remercie.

Je l'ai dit, il s'agit en fait dans toute cette loi de déréguler le travail pour encore plus déformé le partage des richesses et du PIB au profit des actionnaires qui on prélève déjà 10% grâce aux lois précédentes, effectivement de division. Il s'agit. On a parlé de modèle pionnier mais il s'agit enfin de de régime pionnier, il s'agit de casser ce qui pourrait s'en servir aux autres branches c'est le problème du modèle d'une véritable prévention des risques professionnels, prévention. J'ai bien dit et non réparation comme vous le proposerez-vous un peu plus loin. Le mouvement social et les Français sont attachés à leur modèle social, qui ont une autre vision sociétale, dont la réduction du temps de travail et ils sont en train de prendre confiance et de prendre conscience de leur force. Ils avaient ils toutes les tentatives de division qui ont affaibli hier lors de de des réformes précédentes. Mais vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui il n'y a pas de division il y a une unité syndicale et aussi une unité politique de tous les groupes de gauche et des groupes écologistes la division qui a affaibli. Quelques fois les mobilisations hé bien. Vous verrez la semaine prochaine qu'ils vont le dire la semaine prochaine qu'qui ne se laisseront pas diviser. Qui va le dire, tous les Français, les femmes le 8 les jeunes le 9 et le mouvement climatique le 10. Mais. Si. Alors Monsieur Montaugé.

je voudrais dire que on on est vraiment dans une confrontation de 2 modèles de société ce qui oppose. La partie droite de cet hémicycle à sa partie gauche c'était effectivement la vision et la place. Que doivent tenir dans notre vie sociale hein nationale. Les services publics. Toutes les les occasions. Sont saisis par ce gouvernement ou ces gouvernements qui se succèdent depuis quelques années pour affaiblir les services publics et préparer. Je dirais l'avènement total. Des entreprises privées des services privés dans le champ historiquement relevant du service public. En tout cas en France.

Voilà la la meilleure manière de casser tout ça de casser cette forme de pacte social c'était effectivement de remettre en question leur statut. et de préparer l'avènement plus encore que selon le cas aujourd'hui des entreprises privées qui vont rentrer évidemment dans le capital de ce qui reste encore. Dans ce pays. Voilà on l'a on l'a vu avec Gaz de France, Gaz de France n'existe plus. Tout est passé ou quasiment tout est passé au privé avec avec des résultats meilleurs. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que c'est c'est vraiment pas le cas, on le voit, tout particulièrement en ce moment et pour l'électricité, c'est ce qui est en train de se passer

La suppression des régimes spéciaux de retraite est un serpent de mer qui se nourrit évidemment des rancoeurs et des ressentiments et ce n'est pas un hasard si la suppression de certains de ces régimes et discuter dès l'article 1. Toutefois, si le gouvernement joue un jeu dangereux. Je le pense, en opposant les Français entre eux, ils n'en meurs pas moins que la boue mobilisation démontre aujourd'hui que cette stratégie ne fonctionne pas. 9 salariés sur 10 sont opposés à votre projet de réforme. À 64 ans vous n'arrivez pas aujourd'hui à opposer les salariés entre eux. Ils sont côte à côte, qu'ils soient du privé, qu'ils soient du public qu'il soit avec un régime spéciaux ou pas, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez absolument pas à les diviser. Parce que finalement tous ses salariés ce qu'ils ont en commun c'est qu'ils ne veulent pas travailler plus et qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Depuis le début de cet article, hein, vous remettez en cause donc ces régimes spéciaux. Ces régimes que vous qualifiez d'archaïque et que pour nous nous qualifions de. Aujourd'hui d'ailleurs, nous assistons à une perte d'attractivité, ça a été dit autour de ces métiers, il y a un nombre insuffisant de conducteurs à la RATP dans les Hauts-de-France. Il y a eu 100 TER de supprimer. Sur 1200 lignes.

Ticia excusez-moi, vous le savez, l'équilibre est atteint mais vous voulez quand même évidemment leur faire la peau. Ceux et celles que vous applaudissez lors de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, hé bien vous ne pensez plus qu'à ça leur supprimer leur régime et faire en sorte hé bien que demain ces salariés qui sont chaque jour. À nos côtés, hé bien n'est plus leur régime. Merci madame la présidente, mes chers collègues. Monsieur le Ministre vous permettrez. Un membre de la commission des finances de revenir sur l'un des points contenus dans l'article 1, celui de la fermeture du régime autonome de la Banque de France. Je n'en appellerait pas comme tout à l'heure à un illustre prédécesseur Victor Hugo mais une personnalité bien vivante et parfaitement implanté dans notre paysage. Économique, Économique, financier et bancaire. Je veux parler du gouverneur de la Banque de France, monsieur Villeroy de Galhau puisque je l'évoquais tout à l'heure, mais je ne crois pas avoir obtenu la moindre évocation en retour de cette situation et aucun point de vue ni du gouvernement ni des promoteurs de la suppression du régime monsieur Villeroy de Galhau, a exprimé à plusieurs reprises et il vous a écrit. Monsieur le Ministre, le courrier circule dans les services de la Banque de France, il est arrivé juste entre mes mains. Il exprime une forte réticence à l'idée de la fermeture de ce régime. Il rappelle en particulier que. Le régime autonome de la Banque de France a été revu en 2007 avec pour conséquence un alignement total sur celui de la fonction publique il ne comporte donc désormais ce régime aucun Avantage ni privilège ce régime spécial entre guillemets a donc l'unique spécificité d'être totalement financé. Ce qui bien sûr est vertueux, c'est sa seule particularité particularité d'une certaine façon c'est un alignement qui est cohérent puisque les agents titulaires de la Banque de France, recrutés par concours exercent des missions de service public non concurrentiel depuis 2015, la Banque de France a mené une politique non égalé en zone euro. Parmi ses pairs et en France, parmi les acteurs publics de maîtrise de ses coûts avec une baisse de 25% de ses effectifs et une réduction de ses dépenses de 4% par an on volume le maintien du podium autonome. Si la parole Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout à l'heure dans mon intervention j'ai interrogé le ministre-sur le choix qui avait prévalu sur ces cinq régimes. Spéciaux. Je n'ai pas eu de réponse. Je me permets juste d'insister sur le régime spécial des de la RATP en nous renvoyant les uns et les autres à l'actualité qui était celle de notre pays, il y a quelques mois à la rentrée scolaire en particulier. Lorsqu'il y a eu des autorités organisatrices de mobilité en France qui ont été confrontés à une difficulté pour trouver des conducteurs pour le ramassage scolaire et pour le transport scolaire. Dans beaucoup de villes dans beaucoup d'agglomérations dans beaucoup de métropoles. On a dû réduire le nombre de fréquence de passage des bus pour le tout venant pour les rabattre pour le transport scolaire tout simplement ces métiers a été sous tension, comme les métiers dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, je crains fort qu'avec la suppression de ce régime spécial en viennent fragiliser encore plus cette filière et on viendrait fragiliser encore plus ces autorités organisatrices de mobilité qui ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui partout en France. Merci. Alors monsieur le rapporteur. Savary. Oui merci quelques points de précision pour rappeler que jamais nous n'avons parlé. D'inégalités, jamais nous n'avons parlé de privilèges ou de nantis ou même d'archaïsme. Nous avons simplement avec une réflexion approfondie rappeler que il y avait des différences et que ces différences été historique, c'est la raison pour laquelle en contrepartie d'un salaire moins élevé dans nombre de régimes spéciaux, il y avait un départ. Anticipé à la retraite et compte tenu qu'il il était pris en compte justement que ce métier était pénible et ben effectivement leur disait c'est tout à fait légitime. Vous partirez plutôt et en conséquence, la vision de la pénibilité dans ces régimes était vu comme. Une vision réparatrice maintenant on essaye de faire de la prévention et je vois bien que vous êtes impatients de parler de l'usure professionnelle des mesures de prévention qui seront déclinés à l'article 9 et soyez rassurés si nous avançons dans les débats

Il y a eu des pas de fait. Ça fait 4 ans nous que nous parlons de la convergence des régimes spéciaux, nous nous sommes satisfaits de voir que le ministre, le gouvernement nous avait rejoint puisque maintenant on arrive à la fermeture des entrants à travers la clause du grand-père. Et effectivement, ça ne nous avait pas échappé. à travers vos amendements vous proposez maintenant également la fermeture des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Mais ça méritait ni et puis il faut assumer. Nous ça fait 4 ans qu'on assume, vous proposez des dates de fermeture. La date la plus proche, c'est 2027 de fermeture des nouveaux entrants. Nous sommes, nous à 2025 2023 2025. Vous voyez bien j'anticipe sur l'article 7 mai et il faut véritablement assumer cette proposition nouvelle de fermeture des régimes spéciaux, donc pas d'histoire de calendrier entre nous nous règlerons l'affaire à l'article 7. Merci. Alors je vais donner la parole à monsieur le. Président, Laurent, si je suis passé au vote et je voudrais vous demander de vous préparer. Il y aura un scrutin public. merci madame la présidente, moi je veux redire que c'est une grave erreur. Le vote de cet article hein. Il intervient au plus mauvais moment. Vous allez prendre de front si vous votez cette. Les salariés de de secteurs stratégiques, les transports urbains public. Et le secteur de l'énergie, vous allez les prendre de front au moment nous où nous avons à aller où nous Et vous allez créer du chaos dans le pays au lieu. De servir la nation et l'intérêt général. J'ai bien compris, vous allez voter l'article hein mais je voudrais doucher ou décevoir l'enthousiasme du questeur bah qui voit. Un chemin s'ouvrir alors je l'invite le questeur bah à se promener un peu dans les rues de France de Paris le 7 mars prochain et vous verrez que le chemin. Loin de s'ouvrir, va être très très très bouché très très très embouteillés. Parce que vous allez voter ici l'article hein mais ça ne veut pas dire que cette loi va rentrer dans la vie parce que le pays est en train de se lever pour empêcher que cette loi soit adoptée et contre ça, pour le moment vous ne pouvez à rien. Le pays ne veut pas de cette loi. Et la dernière chose que je veux dire c'est. Que. Je voudrais dire au ministre qu'il a pris un risque quand même en donnant son interview au Parisien de demain et on nous on l'a titrée. Je ne sais pas si c'est de l'humour ou si c'est parce que vous cherchez à occuper une place vacante dans le monde des comiques en ce moment, c'est une réforme de gauche. Parce qu'il fallait quand même oser le faire. Alors je veux lui dire qu'il a pris quand même un gros risque en titrant cette interview de cette manière, pas celui de convaincre le pays mais être mardi prochain le la vedette de la risée populaire. Alors je vais donc mettre au au. Donc cet article 1er avec une demande de scrutin public par le groupe socialiste. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 332 pour 233 contre 99, le Sénat a adopté l'article 1er. Alors, mes chers collègues. Je vais lever la séance. Nous avons examiné 300 amendements au cours de la journée. Il en reste 3284 à examiner sur ce texte. Prochaine séance dimanche 5 mars à 9h 30 pour la suite de l'examen du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023. La séance est levée.